Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous à observer, au cours de nos échanges, l'une des valeurs essentielles du Sénat

Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues,

des principes totalement contraires à nos fondements républicains. Ils le font encore en excipant de la belle loi de 1901, c'est-à-dire en recourant au tissu associatif,

troublent le droit de manifester- c'est un droit républicain -, en s'adonnant à des violences parfaitement inadmissibles, que l'unité de la République ne saurait tolérer. monsieur le sénateur, notre conception de l'unité de la République est faite à la fois d'intransigeance et de grande fermeté

Monsieur le Premier ministre, je ne doute pas du tout de vos intentions,

Le creuset de la Nation, de la République, c'est évidemment l'intégration, ce que d'autres appelleraient l'assimilation du passé. C'est cela, créer une Nation qui ait un avenir commun et qui se sente unie dans la difficulté et dans les crises.

tous sont des Français qui servent la République. Monsieur le Premier ministre, faites en sorte que l'État défende la République et la Nation une et indivisible. La parole est à Mme Catherine Fournier,

Tout d'abord, en ce mercredi 9 décembre 2020, jour de deuil national en hommage au Président Valéry Giscard d'Estaing, la famille centriste salue l'action réformatrice de ce grand homme d'État. L'Union européenne faisait partie de l'ADN du Président Valéry Giscard d'Estaing, dont le septennat restera celui de l'instauration du Conseil européen, de la préfiguration de l'euro et de l'élection des eurodéputés au suffrage universel comme en écho, la situation de l'Union européenne est aujourd'hui très préoccupante, puisque, outre la crise sanitaire et la question migratoire, il y a le Brexit. En ce domaine, en lieu et place d'une construction, nous découvrons une destruction ; l'échéance du 2 janvier prochain est imminente, et il n'y a toujours pas d'accord en vue. Passée cette date, c'est l'inconnu pour des milliers de travailleurs et d'entrepreneurs, c'est une inquiétude sourde, que l'élue de la côte d'Opale que je suis ressent singulièrement. La pêche française sera irrémédiablement touchée par un. Sans règle

Monsieur le Premier ministre, les pêcheurs de Boulogne vous l'ont dit, ils vont tout perdre, mais, alors, ils n'auront plus rien à perdre. Demain et vendredi prochain se tient le Conseil européen. La pêche devait être intégrée au paquet global des négociations et, en la séparant du reste, on fait le jeu des Britanniques. Dans ces conditions, la France est-elle toujours disposée à mettre son veto sur l'ensemble des accords si les décisions régissant la pêche ne sont pas satisfaisantes

La question qui est sur toutes les lèvres du pays, depuis quelques jours, est de savoir si la France pourra sortir, le 15 décembre prochain, du second confinement. Vous le savez, le Gouvernement avait fixé comme objectif le seuil de 5 000 nouvelles contaminations par jour. Or nous avons plutôt atteint un plancher de 10 000 nouveaux cas

contre 5 000 par semaine au coeur de l'été. Cette course s'infléchit, grâce à la mobilisation collective des Français ; c'est bien la responsabilité individuelle de chacun qui permet d'alléger la pression pesant sur notre personnel de santé ; il faut le relever et s'en

Nous suivons cela de très près et nous adoptons, en conséquence, les mesures qui s'imposent. Le Premier ministre aura donc l'occasion, demain, en fonction des dernières évolutions constatées et des ultimes arbitrages, de formuler de nouvelles mesures.

toute l'année 2021 ! Oui, il faut informer, mais il faut aussi contrôler les entreprises sur le respect des protocoles sanitaires et il faut supprimer les jours de carence, qui constituent un frein à la prévention pour les salariés du privé. À l'heure où de nombreux Français montrent une défiance à l'égard des vaccins, nous devons sortir de l'emprise du lobby pharmaceutique, en créant un pôle public du médicament. Tel est d'ailleurs le sens de la proposition de notre groupe, que le Sénat doit examiner dans une petite heure. Nous espérons que cette proposition recevra un large soutien. La parole M. Alain Richard, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. nos entreprises et nos services publics se mobilisent et innovent pour y résister et pour remonter la pente, et le plan de relance a commencé à se déployer.

plus de 170 000 aides à l'embauche ont été accordées -, et la qualité des embauches est également à la hauteur des attentes, puisque 70 % de celles-ci sont en CDI. L'apprentissage poursuit également la montée en puissance amorcée depuis le début du quinquennat : nous comptons déjà plus de 420 000 apprentis pour la rentrée de 2020, pulvérisant, si j'ose dire, le record de 2019. Pour apporter une solution à chaque jeune, nous avons également ouvert 300 000 parcours ou contrats d'insertion supplémentaires le 26 novembre dernier, le Premier ministre et moi-même avons encore renforcé le plan Jeunes, afin d'apporter à chaque jeune la possibilité d'un soutien financier, dès lors qu'il s'engage dans un parcours de formation ou dans la recherche d'un emploi. Toute démarche vers l'emploi ou vers la formation mérite

qui s'adresse aux jeunes et aux entreprises et qui vise à faciliter l'orientation, l'entrée en formation, l'emploi et les embauches. Plus de 400 000 jeunes s'y sont déjà connectés, et je sais, mesdames, messieurs les sénateurs, pouvoir compter sur votre mobilisation

La longue liste des données qui pourront être collectées- elle va du parcours professionnel aux habitudes de vie, en passant par les déplacements, les pratiques sportives et la santé psychiatrique -témoigne de cette intrusion dans la vie privée.

C'est le sens de la proposition de loi constitutionnelle que je viens de déposer, en ce jour anniversaire de la loi de 1905, inspirée par mes illustres prédécesseurs radicaux, ceux-là mêmes qui sont aux fondements de notre République. Aujourd'hui, le principe de laïcité se trouve ébranlé par certaines dérives religieuses, mais aussi sectaires et communautaristes. Il était donc temps que soit présenté, ce matin, en conseil des ministres, le projet de loi confortant le respect des principes de la République, afin de nous attaquer aux symboles et d'étayer les murs porteurs que sont nos services publics, nos associations, l'éducation, le sport et la sécurité ; aucun sujet ne doit être tabou. Au rang des avancées, notons le renforcement des contrôles à destination des associations cultuelles masquées en associations culturelles, l'encadrement des fonds provenant de l'étranger, l'effectivité de la neutralité des services publics et la tutelle du milieu sportif ; il était temps, monsieur le Premier ministre, de sortir du déni. En revanche, nous ne serons pas d'accord, vous et moi, sur l'interdiction de l'école à domicile. Si je partage votre objectif d'empêcher certaines dérives, cela passe, à mon sens, par une adaptation des moyens une commission d'entrée et un renforcement du contrôle à domicile, qui ne doit pas incomber aux élus locaux. Le contrôle oui, l'interdiction non ! C'est un contournement d'obstacle qui n'est pas à la hauteur des enjeux.

La laïcité est la liberté de croire ou de ne pas croire, sans contrainte sociale ni étatique. C'est une spécificité française qui fait de nous un modèle dans le monde depuis cent quinze ans. Comment comptez-vous la préserver et l'affirmer dans ce nouveau siècle ? La parole

qui n'est « ni la Bible ni le Coran ». Le nucléaire, avec ses EPR, qui avait été maintenu hors du champ de la Convention, serait maintenant la principale solution. Faut-il comprendre que « le climat, ça commence à bien faire » ? Les coups de com'des engagements d'hier et les coups de gueule d'aujourd'hui sont autant de temps perdu que notre climat ne rattrapera pas. La future loi climat sera tardive son application sera reportée au prochain quinquennat. Encore faut-il qu'elle soit à la hauteur ! Voici ma question : au moment où nous allons, avec l'Union européenne, prendre l'engagement de réduire, non plus de 40 %, mais d'au moins 55 % nos émissions de gaz à effet de serre, comment comptez-vous traduire cela concrètement dans cette loi, alors que les orientations présentées esquivent les propositions les plus fortes ? Y aura-t-il des arbitrages ambitieux sur la rénovation thermique,

à renforcer cette ambition écologique. La France s'est engagée, notamment au travers de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, dans une transition énergétique reposant à la fois sur la sobriété et l'efficacité énergétiques sur la diversification des sources de production et d'approvisionnement, avec le développement des énergies renouvelables. Au travers de la PPE, la France s'inscrit dans une trajectoire. Nous avions besoin de ces repères et de ces objectifs

Sur les trois derniers trimestres, la part des ventes de véhicules électriques a triplé ; le nombre de demandes de MaPrimeRénov'est passé de 10 000 dossiers par mois à 30 000 en octobre

par les liaisons ferroviaires. En effet, nous constatons une réduction excessive du nombre de trains conduisant, dans ce contexte de crise sanitaire, à des situations incompatibles avec le respect de la distanciation sociale. De nombreux trains sont bondés. Quelles mesures le Gouvernement propose-t-il pour veiller à ce que les trains ne deviennent pas de nouveaux clusters ? Qu'en sera-t-il lors du déconfinement ? Par ailleurs, permettez-moi de vous interroger de nouveau

maintenez-vous tous ces financements ? Par ailleurs, les dysfonctionnements qui caractérisent le quotidien de nombreuses lignes Intercités, dont le POLT et ses 3,5 millions d'usagers, vont-ils enfin diminuer ? Enfin,

des passagers dans les trains à réservation, formation et protection des équipes. Cela dit, les études ont montré que seulement 1 % des clusters concernaient les transports.

et de la santé. À ce propos, il faudrait nous dire, monsieur le Premier ministre, si cette absence répétée est due seulement à une simple bouderie ou, plutôt, à un mépris difficilement acceptable des parlementaires de la Haute Assemblée.

Faire de la stratégie, c'est anticiper. Or, sur la question de l'organisation de ces campagnes de vaccination, je crains que nous ne soyons pas vraiment au point. Alors que nos voisins du Royaume-Uni et d'Allemagne sont bien plus avancés que nous ne le sommes- le Royaume-Uni a déjà commencé à vacciner depuis hier et l'Allemagne a déjà mis en place une logistique forte -, qu'en est-il chez nous ? Où en est-on dans l'approvisionnement et les achats de vaccins, et de quel vaccin s'agit-il ? Qu'est-il prévu pour le conditionnement et la conservation des doses, sachant qu'elles doivent être conservées à des températures très basses ? Comment seront-elles acheminées vers les centres de vaccination et où les Français pourront-ils se faire vacciner ? Quel sera le rôle des médecins généralistes ? Sont-ils simplement avertis de l'implication qui sera la leur dans le dispositif de vaccination ?

Monsieur le sénateur, le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur ce point. Je veux vous assurer que cette campagne vaccinale se prépare, et dans de bonnes conditions. Vous avez soulevé un certain nombre de points importants et légitimes

Les vaccins des groupes Moderna et Pfizer devraient être les premiers à obtenir une autorisation européenne. Il ne nous fallait pas l'attendre pour avancer. La Haute Autorité de santé a, ainsi, donné un avis précis sur la stratégie vaccinale,

de transparence. Des questions complémentaires ont, en outre, été transmises à la Haute Autorité de santé, s'agissant, notamment, de l'impact de la sérologie sur la balance entre le bénéfice et les risques individuels de la vaccination. À ce stade, le statut sérologique est neutre sur la priorisation retenue par la Haute Autorité de santé. qui concerne l'acte vaccinal, celui-ci sera, en tout état de cause, réalisé après consultation médicale. Pour la phase 1, un médecin sera présent pour la vaccination, soit pour la réaliser, soit pour la superviser. Il est possible que la question de l'élargissement à d'autres professionnels de santé,

Monsieur le Premier ministre, depuis quelques semaines, la presse, toujours mieux informée que le Parlement, alerte sur les risques que fait peser le projet Hercule sur le service public de l'électricité et sur l'indépendance énergétique du pays. Malgré les interpellations de nos collègues députés, hier, les réponses de Mme Abba ne nous ont guère éclairés. Pourtant, les inquiétudes sont nombreuses, de la part tant des salariés d'EDF, qui craignent de perdre leur statut, que des usagers, du fait du risque d'inflation sur les prix, et des élus locaux. Il est temps d'apporter des réponses à la représentation nationale, que vous ne pouvez ignorer plus longtemps. Nous ne pouvons pas accepter que l'Élysée brade des biens stratégiques dans le dos de la France, pour satisfaire la doctrine libérale de Bruxelles. Il est temps de mettre un terme au démantèlement méthodique de ce fleuron de l'énergie, symbole de la réussite à la française. Il est temps d'arrêter ce processus de libéralisation. Hercule vise clairement le démembrement d'EDF en trois entités. Qu'elles soient « bleue », « verte », « azur » ou autre, les couleurs signent la désintégration totale d'EDF, dans le but inavoué de nationaliser les pertes- c'est-à-dire le nucléaire -et de privatiser les profits autour des énergies renouvelables, les ENR, et de la distribution opérée par Enedis. Il est temps de mettre un frein à la privatisation des barrages en pleine phase de transition énergétique. La France sera le seul pays européen à affaiblir un secteur aussi vital et rentable

Monsieur le Premier ministre, c'est vous que nous voulons entendre, car c'est un sujet de souveraineté nationale. Quel est, précisément, l'état d'avancement des négociations avec la Commission européenne sur ce sujet ? Au travers de quel véhicule législatif comptez-vous faire adopter ce projet de réorganisation ? Enfin, comment répondez-vous au désarroi des salariés ? La

L'objectif de nos échanges avec la Commission européenne est de permettre à EDF de continuer à être l'un des principaux moteurs de la transition. Néanmoins, nous devons nous assurer que le groupe dispose d'un cadre de régulation adapté ... Adapté à quoi ? ... et de capacités d'investissement accrues, pour participer pleinement à la transition.

Vous le savez, nous sommes actuellement en négociation avec la Commission européenne sur la régulation du nucléaire et de l'hydroélectricité. Nous voulons conserver un groupe intégré permettant à l'entreprise de disposer de toutes ses capacités d'investissement, tout en préservant ses emplois et ses savoir-faire.

Face à la délinquance qui explose, au communautarisme qui gangrène les territoires de la République, ... C'est reparti ... ... aux terroristes qui, au nom d'une idéologie fasciste, assassinent des innocents, face aux Black Blocs qui pillent, cassent et sèment la terreur à chaque manifestation, nous étions très nombreux, parlementaires, maires, policiers et gendarmes, à attendre la publication du Livre blanc de la sécurité intérieure. C'est fait. intérieure, la Loppsi 3, et, certainement, au Beauvau de la sécurité annoncé hier par le Président de la République, que le Sénat demandait depuis la remise au Gouvernement du rapport sur l'état des forces de sécurité intérieure en juin 2018. Comme ce livre blanc l'affirme si justement, les maires sont des acteurs centraux de la sécurité communale. Leur responsabilité ne cesse de croître. Ils sont chargés de la politique de prévention auprès de tous leurs administrés. Avec leur police municipale, ils constituent un véritable réseau d'informateurs des forces de sécurité. Vous le savez parfaitement, monsieur le Premier ministre, le redéploiement de la gendarmerie et de la police dans les communes est une question nationale de toute première importance. Ce livre précise, sommairement, les critères de redéploiement territorial, notamment en se fondant sur le nombre d'habitants. Ces critères sont flous et à aucun moment, j'y insiste, il n'est question du premier élu connecté au terrain. À peine publiée, votre proposition de redéploiement intrigue autant les forces de sécurité que les élus locaux. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner les vrais critères de ce futur redéploiement entre les deux principales forces de sécurité, auquel vous ne pouvez manquer d'associer les maires ? Par Par ailleurs, que comptez-vous concrètement mettre en place pour arrêter les Black Blocs dans leur fureur dévastatrice ?

que ce n'est pas une commission, aussi intéressante soit-elle, qui va définir des critères permettant de savoir où iront les gendarmes et la police. C'est en parfaite osmose avec les élus de tous les territoires de la République que nous travaillerons,

Vous soulevez également la question des Black Blocs, ces individus violents, voyous et casseurs. Nous devons casser la dynamique de la peur qui s'empare des centres-villes et, singulièrement, de l'agglomération parisienne.

Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'État aux affaires européennes. Dans notre inconscient collectif, la montagne et l'hiver riment avec de bons moments passés en famille- c'est d'autant plus vrai à l'occasion des fêtes de Noël

L'annonce brutale de la fermeture des remontées mécaniques et l'absence de date de réouverture laissent tous les acteurs dans l'inquiétude. Nous sentons vraiment la colère monter. On nous a expliqué la nécessité d'une coordination européenne. L'Autriche, la Suisse avec laquelle nous avons des domaines skiables communs, et peut-être d'autres pays laisseront leurs infrastructures ouvertes aux vacanciers, tout comme ils ouvriront leurs restaurants. Monsieur le Premier ministre, ce sera le cas, dès demain, à Genève. On nous a, par ailleurs, rebattu les oreilles sur la nécessité de la différenciation. Nous avons compris : la tour Eiffel rouvrira dans une semaine, quand l'intégralité des remontées mécaniques du pays restera fermée pour une durée indéterminée. En matière de différenciation, on peut vraiment mieux faire et ce n'est pas à celle-ci à laquelle nous pensions ! Monsieur le secrétaire d'État, quelle coordination européenne souhaitez-vous poursuivre désormais ? Quelle vraie différenciation locale pouvez-vous proposer aux acteurs de la montagne ?

parce que les activités de plein air seraient les plus dangereuses, mais parce que nous savons qu'il y a aussi des lieux de rassemblement, qui peuvent être dangereux alors que l'épidémie n'est pas totalement maîtrisée. Nous devons être d'une vigilance particulière. J'aurai l'occasion de revenir sur les mesures d'accompagnement et de soutien à l'activité touristique, mais je veux dire que, si nous rouvrions trop tôt, nous prendrions non seulement un risque sanitaire, mais également un risque

La parole est à Mme Sylviane Noël, pour le groupe Les Républicains. Noël, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, quinze jours après les annonces décriées du Président de la République, le monde de la montagne reste encore dans l'incompréhension face aux remontées mécaniques fermées, alors que la tour Eiffel ou le téléphérique de la Bastille, à Grenoble, rouvriront prochainement leurs portes. De qui se moque-t-on ? Le décret paru ce week-end permettant l'accès aux remontées mécaniques à certains usagers, tels que les licenciés d'une association de la fédération française de ski, a suscité beaucoup d'interrogations : comment mettre en oeuvre concrètement une mesure si discriminatoire, qui créera une grande frustration pour les vacanciers privés de ski, pendant qu'ils verront les membres des clubs locaux s'entraîner ? Au-delà, on peut douter de la viabilité financière d'une telle opération, lorsque l'on sait que le coût du fonctionnement journalier d'une station peut frôler les 45 000 euros. jours des vacances de Noël, nous avons besoin de retrouver de la confiance et de la visibilité, à trois points de vue. Nous avons besoin, tout d'abord, d'une visibilité temporelle : les remontées mécaniques demeurent le seul secteur qui ne bénéficie d'aucune perspective quant à la date de réouverture. Quels sont les critères et les seuils qui détermineront cette date ? d'une visibilité organisationnelle. Vous enjoignez aux maires de sécuriser leur domaine skiable pour permettre la pratique d'autres activités. Or de grandes incertitudes demeurent sur les activités en question, notamment celle des jardins d'enfants situés en front de neige. Il est indispensable de délimiter la responsabilité des maires et de permettre un maximum d'activités dans les meilleures conditions de sécurité possible. enfin, d'une visibilité financière. Là encore, de grandes incertitudes pèsent sur les modalités de compensation des pertes d'activité saisonnière pour des entités qui réalisent leur chiffre d'affaires annuel sur quatre mois seulement. Monsieur le Premier ministre, la saison d'hiver est très courte. Pour bon nombre de stations qui fermeront leurs portes dès le mois de mars, le temps presse. Donnez-nous des réponses !

l'ensemble des acteurs de la filière et de la profession, pour évaluer un certain nombre de mesures. Je puis d'ores et déjà vous dire que des mesures d'accompagnement particulières renforcées sont prévues, avec un dispositif de soutien. Je pense tout d'abord à un dispositif de compensation des charges fixes

des travailleurs pauvres, des retraités, des étudiants sans petit boulot viennent allonger désespérément les files d'attente devant les associations d'aide alimentaire, complètement débordées. La crise sociale est là, partout, sous nos yeux. Nous attendions beaucoup du projet de loi de finances, mais le Gouvernement a obstinément choisi de poursuivre sa politique budgétaire et économique. Vous préférez préserver les intérêts des plus fortunés et des grandes entreprises. Vous refusez de faire contribuer fiscalement les plus aisés, dont l'épargne s'est pourtant considérablement accrue. Vous restez sourds et n'acceptez rien- désespérément rien. Vous refusez d'améliorer la prise en charge du chômage partiel comme d'augmenter le SMIC. Prenez-vous la mesure des choses des choses ? Vous privez les Français non seulement de liberté, mais également de fraternité. Même au sortir de la guerre, le Conseil national de la Résistance avait compris qu'il fallait de grandes réformes sociales. Quand allez-vous comprendre qu'il faut une vraie politique sociale, autre que ces mesures d'urgence décidées au coup par coup et insuffisantes ? Quand allez-vous vous inspirer des départements, qui veulent mettre en place un revenu minimum de base ? Quand allez-vous étendre le RSA aux jeunes de 18 à 25 ans ?

Je pense à l'allocation aux adultes handicapés, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à la revalorisation de la prime d'activité, dont vous avez dû lire, dans le dernier rapport de l'Insee, qu'elle avait permis de diminuer le taux de pauvreté dans notre pays. Je vous rappelle aussi que la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté consacre 8,5 milliards d'euros en faveur des personnes les plus précaires dans notre pays. Nous assurons aussi l'accès à la santé pour tous, sans barrière financière : dès le 1 janvier 2021, sera effectif le dispositif avec un remboursement des frais d'optique, dentaires et auditifs. Le Ségur de la santé consacre 100 millions d'euros chaque année à la lutte contre les inégalités en santé, qui est une autre forme d'inégalité puissante dans notre pays. Nous avons instauré la prise en charge à 100 % de tous les frais de santé

Nous avons dégagé des dizaines de millions d'euros pour assurer la mise à l'abri, l'accès à l'alimentation et la mise à disposition de masques. Je me permets, à cet égard, de saluer le travail réalisé par les associations en ce sens. Enfin, vous le savez, nous mobilisons 6,7 milliards d'euros pour le plan « 1 jeune, 1 solution

Voilà une semaine, deux individus placés en détention provisoire pour leur participation présumée à l'attentat de Nice de 2016 ont, ont, contre toute attente, été libérés pour vice de procédure, en l'absence d'une nouvelle ordonnance de maintien en détention provisoire.

Fort heureusement, ces deux Albanais, parce qu'ils étaient en situation irrégulière, ont été interpellés les jours suivants par nos services de police et assignés à résidence.

La même année, a été libéré un jeune homme accusé d'avoir porté des coups mortels à sa mère. Plus récemment, a été libéré, à Marseille, un membre présumé du narcobanditisme. Toutes ces remises en liberté contraintes sont liées à de malencontreuses erreurs de procédure. Dans une démocratie comme la nôtre, la justice est indépendante, ce qui confère aux magistrats de nombreux pouvoirs. Le corollaire indispensable est qu'ils doivent avoir un régime de responsabilité renforcée. C'est la seule réponse à la défiance dont souffre aujourd'hui la magistrature, discréditée par ces négligences, certes minoritaires, mais insuffisamment sanctionnées.

? Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur

que le garde des sceaux a immédiatement diligenté une enquête auprès de l'inspection générale de la justice pour faire toute la lumière sur cette affaire. Je vous le dis de manière extrêmement claire

Madame la présidente, monsieur le ministre des outre-mer, mes chers collègues, je relaie la question de mon collègue et ami Gérard Poadja. « J'ai mal à mon pays », indique l'intéressé, depuis qu'est évoquée la reprise de l'usine du Sud, qui enflamme la Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois depuis trente ans que les Calédoniens s'affrontent de manière aussi violente sur le terrain, avec des barrages sur lesquels certains participants sont armés. Hier, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a indiqué qu'il poursuivrait « inlassablement le dialogue [ ...] jusqu'à parvenir, avec l'ensemble des acteurs, à une solution négociée. » Monsieur le ministre, les consensus ont été la règle dans le secteur du nickel ces trente dernières années : en 1988, lors des accords de Matignon, permettant aux Kanaks d'accéder à l'économie du nickel en 1998, avec l'accord de Nouméa, en décidant de la construction de l'usine du Nord et en organisant l'entrée des intérêts calédoniens au capital de la société Le Nickel et d'Eramet ; enfin, en 2008, lorsque l'usine du Sud a été acceptée par les populations locales. Notre histoire nous a appris que le consensus ne se décrète pas : il se construit. Dès lors, limiter l'espace du dialogue à la seule offre soutenue par l'État, ce n'est pas construire un consensus. Le risque est de répéter les événements des années 1980. est également la fermeture pure et simple de l'usine du Sud, qui mènerait au chômage près de 3 000 familles. Enfin, le risque est la rupture du dialogue politique entre indépendantistes et non-indépendantistes avant un troisième référendum, avec des conséquences difficiles à prévoir sur la paix civile. Ma question est simple, monsieur le ministre : face à ces risques majeurs, le Gouvernement est-il prêt à ouvrir le champ du dialogue au-delà de l'offre actuelle, afin de construire un projet consensuel de reprise de l'usine du Sud ? La parole

saluer le courage des forces de l'ordre- policiers, gendarmes, gendarmes mobiles ... -, qui, depuis maintenant plusieurs jours, interviennent dans des conditions particulièrement difficiles, mais aussi l'autorité judiciaire, qui a commencé à apporter un certain nombre de réponses ces dernières heures.

Si les événements douloureux que nous avons connus dans les années 1980 sont évidemment marqués à jamais dans nos esprits, la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou l'est tout autant. Le dialogue est l'affaire de chacun. C'est un dialogue à trois, dans lequel nous devons tous avancer. Permettez-moi de rendre compte au Sénat des discussions nocturnes que j'ai pu avoir avec les différents protagonistes de ce dossier, notamment sur la reprise de l'usine dite « du Sud », l'usine Vale. Vous le savez, les gouvernements successifs ont soutenu massivement le nickel de manière globale en Nouvelle-Calédonie, et singulièrement l'usine du Sud. Pour nous, la sauvegarde des 3 000 emplois n'est pas négociable.

après l'examen de la proposition de loi portant création d'un pôle public du médicament et des produits médicaux, nous

La séance est reprise. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

de loi. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en juin dernier, en visite dans l'usine de vaccins de Sanofi à Marcy-L'Étoile, le Président de la République a fait de la souveraineté sanitaire de la France une priorité. ainsi débloqué 200 millions d'euros d'argent public pour « financer des infrastructures de production comme de recherche et de développement ».

Or ces financements se font sans condition de contrôle citoyen sur les coûts de production de recherche et de développement. Pis, ces entreprises versent des milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires tout en menaçant de licencier en France et en Europe. En pleine pandémie et crise économique et sociale, il est indécent que certains en profitent pour faire des profits sur la santé et la vie de millions de personnes. Nous avons besoin de développer des capacités publiques de production et de distribution des traitements et des vaccins à l'échelle française et européenne pour que notre santé ne dépende pas des choix financiers de quelques grandes entreprises. C'est le sens de notre proposition de loi portant création d'un pôle public du médicament et des produits de santé, fruit de longues réflexions, de fructueux échanges et de multiples rencontres. En effet, dès 2006 et le scandale sanitaire du médicament Vioxx de la firme Merck, le président François Autain et les membres du groupe communiste républicain et citoyen avaient proposé la création d'un pôle public du médicament, afin de « poser les bases d'une nouvelle règle du jeu plus respectueuse des objectifs de santé publique et d'assurer un rééquilibrage entre les différents acteurs du médicament : les agences, l'État, les citoyens, les médecins et l'industrie pharmaceutique ». Depuis lors, la proposition a été mise en discussion avec les acteurs syndicaux, les associations, les professionnels de santé et les salariés de l'industrie pharmaceutique. Alors que 2 400 ruptures de médicaments ont été constatées en 2020, l'arrivée de la pandémie de la covid-19 a accéléré la démonstration de l'urgence à extraire les médicaments de la loi du marché, pour répondre aux exigences de santé publique. En d'autres termes, de plus en plus de personnes sont convaincues de la nécessité de placer la santé au-dessus des intérêts financiers. Ce fut le sens de ma question d'actualité du 1 avril dernier au ministre de la santé, face au manque de médicaments, de respirateurs et de masques et à la nécessité de mettre en place un pôle public du médicament fondé sur la réquisition des grands groupes

Nous ne pouvons pas rester totalement dépendants en matière d'accès aux médicaments : nous avons besoin d'autonomie, européenne Si même le Gouvernement envisage de le faire, c'est que l'arrivée de la pandémie, en février-mars 2020, les ruptures de stock de masques médicaux de protection, de respirateurs, de médicaments anticancéreux et, plus récemment, de vaccins contre la grippe ont donné du grain à moudre à notre proposition de loi. L'exigence d'une reprise en main, par l'État, de la production et de la distribution de médicaments a été peu à peu reprise par des acteurs de tous bords, du monde politique comme associatif. Ainsi, le rapport sénatorial de 2018 de nos collègues Daudigny et Decool a repris l'idée d'une production publique de certains médicaments essentiels. En juillet 2020, c'est la députée Dubost qui a proposé la création d'un établissement pharmaceutique capable de produire des médicaments au niveau européen. le secteur associatif, des acteurs aussi divers que l'UFC-Que choisir, France Asso Santé, le Conseil consultatif national d'éthique, la Ligue contre le cancer ou l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament sont favorables à la création d'un pôle public de production et de distribution des médicaments considérés comme essentiels. C'est la démonstration que, face aux pénuries persistantes et à l'actualité sanitaire, le rétablissement de souveraineté de la France s'est imposé comme la solution pour un nombre toujours plus important de personnes. Notre souveraineté sanitaire et notre souveraineté industrielle seront remises en question tant que nous ne serons pas en capacité de produire nous-mêmes des produits aussi essentiels. La France paye les choix politiques de désindustrialisation et les délocalisations de la production des entreprises de médicaments en Asie du Sud-Est : voilà seulement vingt ans,

Nous avons les potentiels pour relancer le mécanisme de réindustrialisation d'une filière française des médicaments essentiels. Il manque une volonté politique et des outils de pilotage publics. La crise sanitaire a mis en évidence la dépendance de la France à une production largement réalisée à l'étranger. Et lorsque le Gouvernement évoque le rapatriement sur notre territoire de la production de médicaments, il ne l'envisage que que pour le paracétamol, alors que les besoins sont beaucoup plus importants. De la même manière, Sanofi envisage de rapatrier en Europe une partie de la fabrication des principes actifs. nous savons que son objectif est non pas de revenir en France, mais d'implanter ses usines en Europe de l'Est, où le coût de la main-d'oeuvre est beaucoup moins élevé que chez nous. Notre proposition de loi pose en creux la question de l'Europe libérale, qui monte les peuples les uns contre les autres, au détriment d'une Europe solidaire, qui nous protège, comme en témoigne l'initiative citoyenne européenne lancée par des dizaines d'organisations politiques, associatives et syndicales à travers toute l'Europe, l'Europe, en faveur d'un accès équitable aux futurs vaccins et traitements qui a commencé le 1 décembre dernier, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Je pense également à la question de la filière française du sang et des médicaments dérivés du plasma dont l'activité est menacée. La construction de la nouvelle usine, située près d'Arras, censée augmenter les capacités de production de médicaments dérivés du plasma devrait relever du périmètre du pôle public du médicament. Les conséquences de la pandémie de covid-19 ont démontré l'urgence de sortir les médicaments et les vaccins du secteur marchand. C'est le sens de notre proposition de loi portant création d'un pôle public de production et de distribution des médicaments et des produits de santé, appuyé par un observatoire citoyen, afin de garantir la transparence des médicaments, et financé par la hausse de la fiscalité des assurances.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte soumis à notre examen part d'un constat que je pense unanimement partagé dans cet hémicycle les choix qui structurent aujourd'hui notre politique du médicament ont fini par nous exposer à un phénomène que nous ne découvrons pas, mais que la crise a puissamment révélé, à savoir les pénuries. Les riches auditions que j'ai menées ont été suivies par de nombreuses collègues de tous les groupes au sein de notre commission des affaires sociales, dont je rappelle au Gouvernement l'implication pionnière en matière de lutte contre les tensions d'approvisionnement. Malgré l'absence d'adoption d'un texte de commission, un consensus s'est fait, non seulement sur le diagnostic, mais aussi sur le remède : là où les acteurs privés échouent à convenablement fournir un bien, que l'on peut indiscutablement qualifier de bien public lorsqu'il s'agit d'un médicament essentiel ou d'un vaccin contre une pandémie mondiale, la puissance publique se doit de prendre son relais. On ne manquera pas de m'opposer que des leviers spécifiques ont déjà été aménagés par le législateur, mais leurs insuffisances ne résistent pas longtemps à l'examen. Je pense tout d'abord aux mesures de stockage votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, prévoient que tout exploitant de médicament doit constituer un stock de sécurité ne pouvant être inférieur à quatre mois de couverture des besoins du marché national. cette jauge de quatre mois, dont le Parlement estimait qu'elle définissait moins un plafond qu'un objectif à atteindre, est ramenée par le Gouvernement à seulement deux mois pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, les MITM, cédant ainsi aux pressions des industriels qui craignent une explosion de leurs coûts. coûts. Surtout, quel effet peut-on réellement attendre de cette mesure lorsque l'on sait, par avance, que son application ne fera l'objet d'aucune forme de contrôle ? En 2020, année dont nous conviendrons unanimement qu'elle connut d'importantes pénuries de médicaments, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, n'a pris qu'une seule sanction financière pour rupture de stock, d'un montant non communiqué, mais dont nous savons qu'il est inférieur à 1 million d'euros. Une autre mesure, emblématique, est celle que le Parlement a votée lors de l'examen du projet de loi instituant l'état d'urgence sanitaire et accordant au Premier ministre le pouvoir de recourir à des réquisitions, ainsi qu'à des limitations de la liberté d'entreprendre, pour tout bien ou service indispensable à la sortie de crise sanitaire et dont l'approvisionnement serait temporairement menacé. Alors que les besoins en curare et autres spécialités de réanimation ont frôlé, au cours de la crise, des niveaux jamais atteints, le Gouvernement a préféré s'approvisionner directement auprès des producteurs, payant le prix fort d'un médicament en tension, plutôt que de recourir au cadre légal qu'il s'était lui-même donné à cet effet. Ces demi-mesures ne suffiront pas à endiguer un phénomène de pénuries qui ne montre aucun signe de fléchissement : l'ANSM devrait recenser en 2020 près de 3 200 signalements de ruptures et tensions d'approvisionnement- un record absolu L'obsession de la rentabilité déséquilibre durablement les capacités d'approvisionnement de notre pays en médicaments essentiels, avec des conséquences désastreuses pour les patients. les médicaments régulièrement exposés à des difficultés d'approvisionnement sont en grande partie des médicaments anciens, peu chers, qui intéressent peu les Big Pharma, et qui sont pourtant indispensables dans la prise en charge des patients. Cette situation perturbe l'exercice des professionnels de santé, qui se trouvent contraints de prendre des décisions susceptibles de causer des pertes de chances pour le patient, notamment la substitution par une autre spécialité, qui parfois n'est pas équivalente dont l'efficacité et les effets secondaires pour le patient sont mal connus, la réduction de la posologie administrée ou encore une administration différée du traitement. Face à cette situation délétère, porteuse de dangers, dont la crise sanitaire nous a pleinement fait prendre la mesure, la proposition formulée par mon groupe d'un pôle public du médicament s'inscrit dans la continuité d'exemples étrangers qui ont, chaque fois qu'un tel modèle a pu être déployé, prouvé leur succès. Je pense notamment à la fondation Oswaldo-Cruz de Rio de Janeiro, que j'ai eu l'honneur de visiter en tant présidente du groupe d'amitié France-Brésil, qui produit, sur demande du ministère fédéral de la santé ou des entités mettant en oeuvre divers programmes sanitaires publics prioritaires, des médicaments essentiels, afin de couvrir les besoins du « système unique de santé » brésilien. Retrouvons notre souveraineté, conquérons la maîtrise publique de la production et de la diffusion du médicament. Sans cette maîtrise, nous nous retrouvons avec des groupes pharmaceutiques tels que Sanofi, qui cesse sa recherche et développement sur des thématiques essentielles et qui ferme des sites de production- douze en dix ans, et 5 000 emplois directs supprimés en France. Je viens d'être alertée de l'annonce du directeur général, hier, qui prévoit 400 suppressions d'emplois l'année prochaine. C'est scandaleux Contrairement à certains doutes dont ont pu faire part mes collègues de la commission, le pôle public que nous appelons de nos voeux n'entend pas faire table rase des circuits et des filières d'approvisionnement existants. Il s'agit simplement d'instituer un nouvel acteur, dont les préoccupations seraient exclusivement tournées vers la santé des patients et dont la mission, limitée à l'approvisionnement et à la distribution des médicaments essentiels en tension, serait complémentaire de celle des industriels. Les auditions que j'ai menées ont confirmé le caractère réalisable d'un tel projet si nous établissons en amont la liste des produits essentiels dont nous anticipons les tensions d'approvisionnement et si nous nous appuyons sur un réseau étendu d'acteurs publics et privés, rien ne s'oppose à ce que l'objectif d'un acteur public du médicament, réactif et centré sur des missions, puisse voir le jour. Je reconnais sans difficulté que le texte soumis par mon groupe à votre vote, bien qu'il soit le fruit d'une réflexion aboutie, entraînerait quelques difficultés d'application, notamment en termes de concurrence de compétences entre le pôle public du médicament que nous créons et les agences sanitaires existantes. Toutefois, si nous partageons l'intention profonde qui anime ce texte, monsieur le secrétaire d'État, il me semble que ces difficultés pourront être facilement levées par la navette parlementaire. Outre la création du pôle public du médicament, la proposition de loi vise un objectif plus large, celui de lutter contre la défiance croissante de nos concitoyennes et concitoyens à l'égard des produits innovants, notamment des vaccins. cette défiance trois causes, qui se nourrissent d'une opacité persistante et entretenue autour des grandes étapes de la vie du produit médical innovant, en amont et en aval de sa commercialisation les financements qui accompagnent la recherche et la participation de l'effort public ; ensuite, la négociation du prix, dont le niveau peut parfois atteindre des chiffres indécents, qui limitent son accès précoce ; enfin, les démarches de pharmacovigilance et de matériovigilance, qui accompagnent la commercialisation. commercialisation. Il est incontestable que règne sur la recherche fondamentale une opacité entretenue par le « secret des affaires nous sommes aujourd'hui dans l'incapacité de chiffrer avec précision non seulement les dépenses consenties par l'État au titre du crédit impôt recherche, le CIR, en soutien aux entreprises privées, mais aussi le prix de cession payé par ces dernières, lorsqu'elles acquièrent un brevet d'invention, largement financé par des organismes publics de recherche. L'article 38 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, que nous avons adopté, constitue un pas en avant, mais qui est encore insuffisant. concerne le prix du médicament ou du produit innovant, il n'est plus admissible que la détresse et l'urgence qu'entraînent certaines maladies rares confèrent aux grands laboratoires le pouvoir léonin d'imposer leur prix, à charge pour les régimes sociaux de s'y conformer. Certains d'entre vous ont peut-être en mémoire l'exemple malheureux du Zolgensma, ce médicament de thérapie génique destiné à soigner une maladie dégénérative très rare frappant les nouveau-nés, pour lequel le laboratoire Novartis demandait à l'assurance maladie une indemnité de 2 millions d'euros par unité ! Face à des industriels pharmaceutiques de grande taille, dont les marchés dépassent très largement le territoire national, et privés de connaissance sur les coûts réels de production des médicaments innovants, nous nous retrouvons contraints, pour fournir ces précieux produits à nos concitoyennes et concitoyens, de signer le chèque. Ainsi, il paraît aussi souhaitable que réalisable que la fixation du prix du médicament innovant intègre, aux côtés du critère principal de l'amélioration du service médical rendu, d'autres critères permettant d'objectiver sa valeur économique réelle et de permettre que son coût pour les finances publiques soit rationalisé et mieux accepté. les grands scandales sanitaires de notre époque, dont celui du Mediator demeure le plus probant exemple, nous imposent de renforcer la vigilance portée aux produits innovants qui ont fait l'objet d'une commercialisation. Encore inaboutie, bien qu'elle soit en progrès pour les médicaments, cette vigilance continue de présenter d'alarmantes lacunes pour les dispositifs médicaux, relayées par le rapport récent de nos collègues députés Julien Borowczyk et Pierre Dharréville. À cet égard, l'article 4 de ce texte propose la mise en place d'un observatoire citoyen des vigilances, placé auprès de l'ANSM, mais totalement indépendant, chargé de vérifier la transparence des signalements d'événements indésirables. n'attendons pas simplement qu'un nouveau scandale et de nouvelles victimes nous ouvrent brutalement les yeux sur des défaillances d'un système dans lequel nos concitoyennes et concitoyens, atteints de pathologies, placent légitimement leur confiance. Dotons-nous, dès aujourd'hui, des instances nécessaires à déclencher les alertes pour renforcer notre démocratie sanitaire. Des fissures, voire des fractures, marquent chaque jour un peu plus notre modèle social. Nous portons ici la voix des oubliés, des vulnérables, de toutes les personnes blessées par une mondialisation sauvage et une course au profit qui n'épargnent plus le seul bien dont nous pensions nous enorgueillir de ne pas l'avoir mis à vendre : la santé.

prend un sens tout particulier dans la période que nous connaissons, où il n'a jamais été autant question de l'accès aux médicaments. La crise du covid-19 a révélé, ou plus exactement confirmé, les fragilités et les difficultés de la chaîne d'approvisionnement. Je dis bien « confirmé », parce que cela fait plusieurs années, malheureusement, que nos concitoyens et les professionnels de santé qui les soignent sont confrontés à des ruptures de médicaments. Les chiffres sont là les signalements de ruptures de stocks et de tensions d'approvisionnement ont été multipliés par vingt entre 2008 et 2018, quelque 80 % des principes actifs pharmaceutiques sont fabriqués hors de l'Union européenne, principalement en Chine et en Inde, et 40 % des médicaments finis commercialisés dans l'Union sont en provenance de pays tiers. Ces chiffres, dont vous avez rappelé quelques-uns, madame la sénatrice, ne sont pas une fatalité, bien au contraire. Ils doivent constituer un levier pour avancer vers une plus grande autonomie stratégique au niveau européen.

La relocalisation de la production pharmaceutique au sein de l'Union européenne et l'innovation dans ce domaine, conformément aux objectifs du, sont la condition et la garantie d'une autonomie stratégique européenne.

intitulée, construite autour de vingt-huit actions regroupées en quatre axes, dont le renforcement de la coopération européenne. Nous poursuivrons donc, dans les prochains mois, les actions entreprises, en soutenant notamment la mise en place de la stratégie pharmaceutique pour l'Europe, présentée le 26 novembre dernier, par la commissaire européenne à la santé Stella Kyriakides. Cette stratégie devrait permettre à l'Union européenne de tendre vers davantage de souveraineté sanitaire et d'investir avec pertinence dans la recherche. Dans ce cadre, il est notamment prévu de créer une nouvelle instance pharmaceutique, l'Autorité européenne d'intervention en cas d'urgence sanitaire, pour faire face aux attentes médicales et urgences pharmaceutiques. Il est également prévu de renforcer la présence de l'Union européenne à l'échelon mondial, en mettant en place des règles égales pour tous les acteurs du secteur et à toutes les étapes du médicament- de la recherche à l'autorisation, de la consommation à la fin de vie de ces produits. les sénateurs, nous sommes convaincus qu'une partie de la réponse de demain est européenne. Mais, sans attendre, ce sont bien des mesures nationales que nous avons prises pour soutenir la diversification de la chaîne d'approvisionnement et augmenter la capacité de production en France. Dans ce contexte, nous avons adapté notre action avec le plan de relance, pour accélérer ces transitions et pour construire, dès aujourd'hui, notre souveraineté sanitaire et industrielle. Nous mobilisons au total 100 milliards d'euros, dont près de 35 milliards d'euros pour l'industrie. Le volet industriel de ce plan repose sur quatre piliers : améliorer notre compétitivité pour localiser davantage d'activités en France ; faire de la transition écologique un avantage comparatif moderniser notre appareil de production ; innover pour nous positionner sur des marchés d'avenir. Le secteur de l'industrie médicale va bien évidemment bénéficier du plan de relance : 6 milliards d'euros seront investis dans les infrastructures médicales et plus de 20 milliards d'euros dans la recherche et dans l'innovation. En parallèle de ces actions en faveur de la réindustrialisation, nous nous sommes également dotés, sur le plan national, de mesures réglementaires pour résoudre le problème de la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement. Il s'agit d'actions que vous connaissez pour les avoir examinées lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Je pense notamment à la création d'une obligation pour l'industrie pharmaceutique de constituer des stocks de médicaments destinés au marché national. Le projet de décret pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale votée en 2019 a été transmis au Conseil d'État et se trouve en cours de notification à la Commission européenne. Enfin, les sanctions financières ont également été renforcées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, ce qui permet à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de disposer de nouveaux motifs de sanctions financières en cas de non-respect des obligations incombant aux entreprises.

». Nous partageons certains de vos constats ; pas tous, vous vous en douterez. Nous partageons même l'idée selon laquelle la question d'un programme public de production pourrait faire sens. Nous avions d'ailleurs inscrit, dès 2019, au travers de l'action n° 20 de la feuille de route ministérielle que j'évoquais à l'instant, la nécessité d'expertiser la mise en place d'une solution publique pour organiser des approvisionnements en cas de pénurie. les propositions que vous formulez ne nous semblent pas prendre en considération toutes les dimensions du problème. Tout d'abord, plusieurs acteurs publics, dont Santé publique France, disposent déjà de prérogatives concernant l'importation, l'acquisition groupée ou la distribution de produits de santé, ce qui s'est traduit très concrètement dans le cadre de la prise en charge des patients covid-19, notamment lors de la régulation nationale pour deux hypnotiques et trois curares. Ensuite, nous sommes convaincus que la diversité des acteurs, publics et privés, français et étrangers, est nécessaire pour assurer l'approvisionnement des populations en produits de santé, pour maintenir un haut niveau de qualité des produits et pour favoriser le développement de l'innovation. C'est là où la création d'un programme public isolé du reste du paysage industriel atteindrait certaines limites opérationnelles. Quels seraient les médicaments concernés ? Pour quel marché ? Selon quel modèle économique ? Pour conclure, mesdames, messieurs les sénateurs, et faire écho avec le début de mon propos, fonctionner selon une approche franco-française n'aurait pas vraiment de sens, et surtout ne permettrait pas de mettre en place un outil productif viable, seul à même de garantir la sécurité des patients dans le long terme. C'est bien au niveau européen que la réflexion doit être menée sur l'opportunité de créer un ou plusieurs établissements d'intérêt public à but non lucratif, dont l'une des missions serait particulièrement adaptée à la production de médicaments matures, essentiels et indispensables pour certaines prises en charge.

La crise du covid a provoqué un déclic, et il n'est plus aujourd'hui avant-gardiste de parler de résilience industrielle européenne. La France et ses industries doivent être les fers de lance de cette souveraineté, et nous devons porter des projets communs au plan européen. En effet, face à certains marchés dynamiques et historiques, nous ne ferons le poids que si nous construisons un écosystème industriel européen concret. La parole

et nous ne désespérons pas de voir émerger à court terme des solutions concrètes, susceptibles de mettre fin à la situation dramatique que nous connaissons. Cette situation, c'est une tension qui ne fait que croître de manière exponentielle depuis quelques années. Ce sont 404 médicaments signalés en rupture ou en risque de rupture en 2013, puis 1 500 en 2019 et déjà 2 400 pour 2020, soit six fois plus qu'en 2013. Ces chiffres, nous ne cessons de les répéter, comme nous le rappelle le rapport de nos collègues Daudigny et Decool, dont les trente propositions ont conduit à la rédaction d'une proposition de loi que nous sommes nombreux à avoir cosignée.

Les tensions d'approvisionnement sur les médicaments entraînent en effet des pertes de chances importantes pour les patients, sans compter le temps que doivent désormais y consacrer les professionnels de santé. On parle de 16 équivalents temps plein rien que pour l'AP-HP. Ces tensions concernent en grande partie des produits matures et peu coûteux, mais aussi des médicaments anticancéreux, antibiotiques et antiparkinsoniens, essentiels pour les patients. Il est inutile de rappeler les conséquences la pénurie en anesthésiants au début de l'épidémie de covid, ni celle du vaccin contre la grippe cet automne. Les industriels proposent jusqu'ici des solutions qui ne sont pas satisfaisantes et sont incapables de répondre aux fluctuations, même attendues, de la demande. Or il s'agit pour notre pays d'une question de souveraineté dans un domaine stratégique, je dirais même vital.

On ne peut pas dire que rien n'a été fait dans le domaine. Des actions ont été entreprises depuis 2016 par les gouvernements successifs : mesures de prévention et de gestion des ruptures de stock dans la loi de 2016, possibilité pour les pharmaciens de remplacer un médicament en rupture par un autre depuis 2019, plan de gestion pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et, bien sûr, la feuille de route 2019-2022 pour lutter contre les pénuries, dont les effets tardent à se faire sentir et dont nous attendons l'évaluation annuelle, telle qu'elle est inscrite à l'action n° 28. En juin dernier, face à l'aggravation de la situation, le Gouvernement a présenté un plan d'action pour agir sur la relocalisation de sites de production de produits de santé, car c'est bien de cela qu'il s'agit dans la proposition de loi que nous examinons. C'est dans ce sens qu'il faut aller, mais dans le cadre d'une réflexion plus globale et d'une action coordonnée. En effet, les tensions d'approvisionnement ont des origines multifactorielles, tout au long de la chaîne de production et de distribution, et ne sauraient être résolues par une solution unique. La proposition de loi prévoit cinq actions, dont certaines suscitent de notre part certaines réserves. Si nous sommes tout à fait favorables au renforcement de la transparence, de la démocratie sanitaire et de l'éthique nous sommes plus mesurés sur la création d'un pôle public du médicament et des produits médicaux, financé par une hausse de la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques. Nous doutons tout d'abord que cette hausse de taxe suffise à elle seule à financer une telle mesure. Nous craignons ensuite qu'elle ne vienne accentuer les délocalisations, en poussant les entreprises à fuir davantage notre pays. C'est un modèle de nationalisation que, à titre personnel, je ne partage pas. Surtout, ce qui manque à cette proposition de loi, c'est la dimension européenne, qui est intrinsèquement liée à la question des pénuries de médicaments et de vaccins. Nous ne pouvons agir seuls sur ce sujet. Le Gouvernement a pleinement identifié ce point, en travaillant à une coordination européenne pour renforcer notre autonomie stratégique en matière de santé et mieux faire face aux crises sanitaires. La commande groupée de vaccins contre la covid est une première étape indispensable, avant, je l'espère, la construction d'une véritable Europe de la santé, que nous appelons de nos voeux. Toutefois, il aura fallu une crise sans précédent et plus de 50 000 morts en France pour faire bouger les lignes.

S'agissant de la proposition de loi, si, sur le fond, notre groupe en partage l'analyse, nous doutons davantage de la faisabilité et de l'efficacité de la solution proposée.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, « tant qu'on a essayé de combattre la peste avec des mots latins, elle a tranquillement dévoré l'humanité » a écrit Barjavel. Nous sommes d'accord, face à la maladie, nul besoin de longs discours. Il faut des substances actives thérapeutiques. Dans un contexte de pandémie mondiale, ce constat prend une résonnance particulière. Or, précisément, pour le patient en puissance qu'est chacun de nous, accéder à un traitement ne va plus de soi. Le risque est grand, parce que les médicaments sont des produits « ultra-essentiels », parfois vitaux, et parce que la nature a horreur du vide, de voir s'organiser des marchés parallèles plaçant les acheteurs dans une situation de vulnérabilité particulièrement préjudiciable. Pour pallier ces difficultés, notre collègue Laurence Cohen et son groupe nous proposent aujourd'hui la création d'un « pôle public du médicament et des produits médicaux ». De juillet à septembre 2018, nous avons participé, sous la présidence d'Yves Daudigny, à la mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins.

Même si le contexte est exacerbé, le problème n'est pas nouveau. Les tensions d'approvisionnement se confirment, hélas, depuis quelques années, et les effets de ces pénuries sont de plus en plus pénalisants pour les patients. En fait, c'est toute la circulation mondiale des produits de santé qui est en cause, et la France en fait les frais. Le non-accès du patient à un médicament ou sa non-délivrance par le pharmacien est une situation insupportable et inacceptable, tant pour le malade que pour le professionnel de santé. Ces situations, au-delà même du risque de perte de chance, sont anxiogènes et chronophages, dans un pays où, par ailleurs, l'on manque de temps médical. Une telle situation

Il est important de le préciser, une « rupture d'approvisionnement de médicaments » est une situation précise, définie par les termes du décret du 28 septembre 2012, qui est caractérisée lorsqu'« une pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur est dans l'incapacité de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures ». Cette rupture d'approvisionnement peut être imputable, notamment, à une rupture de stock ou à une rupture dans la chaîne de distribution. Il est important d'avoir des définitions homogènes. Nous touchons du doigt la complexité d'une chaîne qui agrège plusieurs acteurs, chacun des maillons se trouvant dépendant du maillon antérieur et chaque liaison constituant un potentiel point de rupture. Une première difficulté réside dans l'absence de visibilité sur la durée du manque. En effet, au-delà de 72 heures, on peut se trouver dans un délai de réapprovisionnement de quelques jours, quelques semaines ou plusieurs mois, et la stratégie de rechange à mettre en place dépend directement de cette indispensable visibilité. J'écarte le sujet des « microruptures » de moins de 72 heures, qui échappent aux comptages, mais polluent la vie des malades et soignants. J'ai bien noté, aux articles 2 et 4, votre souhait de travailler à apporter plus de transparence. Actuellement, les outils d'information sont améliorables. Il est d'ailleurs prévu dans la feuille de route 2019-2022 d'élargir la plateforme DP-Ruptures à toute la chaîne de distribution, incluant grossistes, répartiteurs et dépositaires, dans le cadre d'un outil partagé de signalement. Le sujet est d'autant plus complexe que les causes de rupture d'approvisionnement sont nombreuses et multifactorielles. Les difficultés sont d'abord liées à la production : capacité de production insuffisante, retard de production, incapacité de production par manque de matières premières, responsable de 17 % des ruptures,

les évolutions du marché du médicament, avec l'éclatement des différentes étapes de fabrication pour optimiser les coûts - je pense aux lignes de production programmées par périodes -, la recherche d'une rentabilité à court terme, qui a notamment conduit à travailler à flux tendus, sans stocks et, enfin, le développement des marchés émergents. en cas de rupture d'approvisionnement anticipée ou constatée, qui fait quoi ? La loi du 29 décembre 2011, relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé,

que le soin soit indissociablement soumis aux contraintes de la loi du marché. Vous proposez de sortir les médicaments du marché, au moins partiellement. Est-ce possible ? Est-ce la solution ? En relisant nos débats et les auditions de 2018, avant même la crise sanitaire, vous en faites d'ailleurs état vous-même, vous aviez déjà, chère collègue, l'idée d'un laboratoire public du médicament. Voici la réponse Voici la réponse que vous avait adressée l'une des sous-directrices de la direction générale de l'offre de soins : « L'intérêt de l'État est plutôt de renforcer son rôle de régulateur et de coordonnateur entre autorités compétentes que de développer un rôle d'industriel où il pourrait se retrouver en difficulté au sein d'un marché très concurrentiel. Vous avez mené un travail de fond considérable, mais je ne partage pas vos conclusions. En effet, un pôle public de production et de distribution de médicaments pourrait-il régler le problème de l'accès aux matières premières ? Si ce pôle concentre son activité sur la production de médicaments devenus non rentables, alors l'État supportera la charge financière d'une production à perte. Y a-t-il un chiffrage à cet Quelles solutions envisager pour les problèmes de logistique et de stockage, car la fragilité n'est pas concentrée au niveau de la production ? Enfin, l'article 5, qui vise à taxer l'industrie pharmaceutique, semble plutôt dissuasif et contraire à une dynamique de relocalisation. Si l'intention de ce texte est louable, et si nous partageons l'objectif d'accès au médicament en tout temps, en tout lieu et pour tous, il ne nous semble pas être de nature à permettre d'éviter réellement les pénuries de médicaments. Face à des difficultés qui deviennent structurelles, peut-être faudrait-il plutôt envisager une réforme de la politique des prix du médicament, qui sont devenus, au fil des PLFSS successifs, une variable d'ajustement,

Ne serait-il pas pertinent de travailler à la constitution de stocks suffisants pour répondre aux besoins des usagers, tout en veillant à ne pas engager une tendance mondiale au stockage, ce qui « assècherait » la ressource et constituerait un facteur de pénurie ? Pourquoi ne pas renforcer dans la loi et dans les faits les sanctions envers les laboratoires négligents dans l'approvisionnement du marché français ? travailler à des appels d'offres par segments spécialisés, avec plusieurs attributaires ? La réflexion doit se poursuivre. Parallèlement, il est prudent d'attendre, afin d'évaluer les effets de la feuille de route 2019-2022 en cours

la pandémie de la covid-19, qui a endeuillé notre pays, l'Europe et le monde, a fait ressurgir dans le débat public les difficultés et les faiblesses de la France et de toute l'Europe dans le secteur du médicament. C'est l'échec des stratégies de rationalisation qui sont choisies par les grands laboratoires pharmaceutiques et acceptées et subies par notre système de santé. Plusieurs d'entre vous l'ont dit, cette situation n'est pas nouvelle, et je tiens à remercier Laurence Cohen et l'ensemble du groupe CRCE d'avoir, par cette proposition de loi, permis de revenir, dans cette assemblée, sur cette question majeure. Nous partageons les constats dressés par Laurence Cohen dans sa proposition de loi, notamment la nécessité d'une solution publique de production. de production. Aujourd'hui, près de 40 % des médicaments finis commercialisés dans l'Union européenne proviennent de pays tiers, et 80 % des fabricants de substances pharmaceutiques actives utilisées pour des médicaments disponibles en Europe sont situés en dehors de l'Union, contre 20 % seulement voilà trente ans. Les politiques ultralibérales et la course aux dividendes démontrent une fois encore leurs effets néfastes. Cette délocalisation croissante est l'une des causes des pénuries de médicaments à intérêt thérapeutique majeur en France. Encore marginal avant les années 2010, avec seulement 44 ruptures de stock en 2008, le nombre de pénuries de médicaments ne cesse de croître depuis le début de la décennie. En 2019, on en recensait 1 200, et l'ANSM envisage leur doublement en 2020. Ainsi, 2 400 médicaments devraient être touchés. Le débat parlementaire dans le cadre de l'examen du PLFSS 2021 a d'ailleurs été largement marqué par la question des pénuries de médicaments. Notre groupe avait pris toute sa part, avec des propositions fortes, telles que l'obligation d'un stock de sécurité de quatre mois, pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur. ait été adopté par le Sénat, l'amendement en question a été supprimé par la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale, ce que nous ne pouvons que déplorer. Autre constat partagé, le défaut de transparence dans le domaine du médicament. La crise du coronavirus a mis en lumière le rôle majeur joué depuis toujours par la puissance publique dans le financement de la recherche et développement dans le domaine de la santé. Or les sommes investies par l'État ne sont jamais rendues publiques et ne sont pas prises en compte dans la négociation des prix des produits de santé avec les entreprises pharmaceutiques. Nous ne pouvons que le constater, les pouvoirs publics règlent deux fois l'addition. Dans un premier temps, l'État finance les investissements de recherche et développement non seulement dans le public, mais aussi dans le privé, au travers notamment du crédit d'impôt recherche. Dans un second temps, l'assurance maladie supporte, sur le long terme, le coût de l'innovation, du fait des mécanismes de fixation des prix. Le Comité économique des produits de santé, le CEPS, n'ayant pas connaissance des investissements publics ayant participé au développement d'un médicament, la question de la transparence se pose. Les négociations, vous le savez, sont secrètes. Face à ces situations, force est de constater que les gouvernements n'ont fait que de la gestion de crise. Or c'est toute une politique en matière de souveraineté et de sécurité dans le domaine de la santé qui est à revoir. Le manque de démocratie sanitaire et de transparence dans les prises de décisions politiques sanitaires est aussi à regretter et à condamner. La crise du covid-19 en est d'ailleurs un parfait exemple. Ni les citoyens, ni les élus locaux, ni même les associations d'usagers du système de santé n'ont été pleinement associés à la gestion de la crise. Il convient donc, dès à présent, de renforcer notre démocratie sanitaire, notamment au moment où nous allons entrer dans une campagne de vaccination contre la covid-19. Dans cette philosophie, nous soutenons la nécessité de renforcer l'implication citoyenne dans la surveillance des médicaments et des dispositifs médicaux après leur commercialisation par la création d'un observatoire citoyen. Nous défendrons un amendement sur ce point. L'industrie pharmaceutique étant constituée essentiellement de laboratoires multinationaux, les Big Pharma, la France ne peut agir seule. Une coordination avec les États européens est indispensable. L'Union européenne est d'ailleurs en train de renforcer sa politique de la santé et du médicament. Pour la première fois, l'Europe, qui ne dispose que d'une compétence d'appui centrée sur la coordination des actions des États membres, a été en mesure de passer des « commandes groupées » de futurs vaccins en cours d'expérimentation, pour ses pays membres. Par ailleurs, dans le cadre d'une plus grande implication de l'échelon européen dans la stratégie de santé pour faire face à la crise sanitaire, le 11 novembre dernier, la Commission européenne a prévu d'accroître le rôle du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de l'Agence européenne des médicaments. Elle envisage de la doter d'effectifs et de moyens supplémentaires, afin qu'elle puisse davantage surveiller les stocks de matériel médical et de médicaments et prévenir des risques de pénurie.

Enfin, la Commission européenne envisage la création d'une nouvelle autorité en 2023 pour une meilleure coordination face aux menaces sanitaires transfrontalières. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat partage l'ensemble des constats dressés par Laurence Cohen dans sa proposition de loi. Nous pensons, nous aussi, qu'une reprise en main de la politique du médicament et de la santé par les pouvoirs publics est indispensable. La France doit retrouver sa souveraineté en matière de santé et faire passer les intérêts de ses concitoyens avant les intérêts particuliers des grands laboratoires pharmaceutiques.

la France dispose de moyens déjà existants pour produire les médicaments sujets aux défauts d'approvisionnement. L'Agence générale des équipements et produits de santé, l'Ageps, et la pharmacie centrale des armées, deux laboratoires publics, sont susceptibles de pouvoir produire des médicaments. Ainsi, en 2009, lors de la crise de la grippe HIN1, la pharmacie centrale des armées avait produit 77 millions de comprimés de Tamiflu. de Tamiflu. Le dispositif de la licence d'office existe également, au cas où l'intérêt de la santé publique serait menacé par un approvisionnement insuffisant de spécialités pharmaceutiques. Il permet de contraindre le titulaire du brevet d'un médicament à autoriser l'exploitation de son brevet par des tiers et de manière non exclusive. Néanmoins, peut-être la volonté politique fait-elle défaut pour activer ces leviers. Leur exploitation est aujourd'hui insuffisante et mal adaptée aux enjeux. Il nous semble qu'une meilleure coordination avec les organismes existants permettrait de répondre plus efficacement et nationalement aux besoins de médicaments de nos concitoyens en période de crise et de pénurie.

Il y va non seulement de la réindustrialisation de notre pays, source d'emplois et de richesses pour nos territoires, mais aussi, et surtout, de notre souveraineté et de notre indépendance. Ce qui paraissait utopique et inimaginable il y a peu de temps paraît aujourd'hui réalisable.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le temps des tempêtes est toujours propice à la mise en lumière des carences, des faiblesses et des errements collectivement commis. La pandémie du coronavirus n'a pas échappé à ce phénomène et a révélé les errements du monde qui s'est construit sous nos yeux un peu coupables depuis plusieurs décennies. Qui aurait pensé que nous manquerions de médicaments aussi basiques et nécessaires que le paracétamol ? Pénuries, absence de coordinations entre chaînes de productions et de distributions, asphyxie des services de santé : la liste est longue, et nous la connaissons tous. il faut toujours une prise de conscience douloureuse pour se pencher sur certains enjeux jusque-là sous-estimés. L'indisponibilité des médicaments et des vaccins est aujourd'hui chronique. Elle concerne l'ensemble de ces produits. Durant ces années de mondialisation incontrôlée, nous avons progressivement perdu notre souveraineté sanitaire, au profit de puissances étrangères non européennes. Les chaînes de production s'en sont retrouvées éclatées à l'autre bout du monde, alors que, dans le même temps, la forte hausse de la demande mondiale suscitait des concurrences délétères dans l'approvisionnement en médicaments. La reconquête industrielle et sanitaire doit être un tournant : elle doit en effet nous conduire à changer le paradigme qui nous a menés dans l'impasse. Comment accepter sans rien dire, au sortir de la crise de la covid, les déclarations de Paul Hudson, qui déclarait que Sanofi servirait « en premier » les États-Unis s'il trouvait un vaccin ? Doit-on considérer les produits de santé indéfiniment soumis à la loi du marché mondialisé ? Il nous faut donc impérativement enclencher tous les leviers, qu'ils soient Français ou européens. Il convient relocaliser l'industrie pharmaceutique, deuxièmement, d'engager une démarche de clarté dans la gestion des stocks et des commercialisations par les groupes pharmaceutiques, de planifier et d'organiser, dans l'esprit interventionniste d'un État stratège, les politiques publiques de production, tarification et distribution de certains médicaments, en temps de crise comme en période plus calme. Madame la rapporteure, votre proposition de loi a le mérite, je l'ai dit, de poser le grave problème de la souveraineté sanitaire. Elle mérite, j'en suis intimement convaincue, que nous en débattions et échangions en révisant certains logiciels et paradigmes idéologiques qui ont fait mal, ces dernières années, à la fois à notre système de santé et à notre tissu industriel. Pour faire face à cette pénurie, vous proposez la création d'un pôle public du médicament.

Les différences de prix pèsent également sur les stratégies d'allocation des stocks par les laboratoires. S'agissant de la création d'un pôle public du médicament, fait l'objet de l'article 2 de votre proposition de loi, l'idée peut être séduisante. Encore faudrait-il concevoir une structure opérationnelle, sur les plans tant de son financement que de son organisation.

doute, monsieur le secrétaire d'État, pourriez-vous nous préciser l'état de la mise en application de ce texte ? L'État stratège, c'est aussi un État qui crée une véritable stratégie industrielle nationale et européenne, pour engendrer les conditions d'une production pharmaceutique de proximité. Nous pourrions envisager un panel d'incitations, en contrepartie d'engagements prévus dans un accord-cadre liant les industriels et l'État. Le pôle public du médicament dont vous proposez la création pourrait alors se concentrer sur la production et la distribution de médicaments « de niche », régulièrement exposés à des tensions d'approvisionnement. C'est là que la pharmacie centrale des armées et l'Agence générale des équipements et produits de santé pourraient intervenir. En revanche, en ce qui concerne la réquisition des laboratoires pharmaceutiques en temps de crise, il paraît selon nous difficile de rendre l'entreprise responsable d'une problématique qu'elle ne maîtrise pas complètement, à savoir le cycle production-commercialisation. Madame la rapporteure, mes chers collègues, la pandémie a mis à mal certains clichés : depuis la crise, les termes de « souveraineté » et d'« indépendance » ne sont plus des gros mots, même dans les chapelles du nouveau monde- c'est peu dire La souveraineté, c'est notre capacité à déployer plusieurs solutions face à un problème multifactoriel. Il ne suffit pas, en effet, de décréter l'autonomie pour qu'elle se réalise. C'est en cela, madame la rapporteure, que je juge votre texte bien intentionné, mais non abouti. Nous ne pouvons le suivre. Avant de vouloir densifier le système actuel en le dotant d'une institution supplémentaire,

nous devons avant tout nous poser la question de l'efficacité de la mesure. Mes chers collègues, cette proposition de loi a le mérite de poser, une nouvelle fois, la question de notre souveraineté sanitaire.

le plus grand producteur au monde de vaccins : le. Ces 60 millions de doses devraient permettre, selon les protocoles sélectionnés, de vacciner entre 25 et 32 millions de personnes.

Je n'entrerai pas dans la polémique sur la course de vitesse engagée par les laboratoires, mais cet exemple illustre parfaitement le décrochage de l'industrie pharmaceutique française et européenne. Les unités de fabrication de médicaments et de vaccins sont désormais quasiment le monopole de l'Asie. Nos sites se sont exilés. Selon l'Agence européenne du médicament, « près de 40 % des médicaments finis commercialisés dans l'Union européenne proviennent de pays tiers, et 80 % des fabricants de substances pharmaceutiques actives utilisées pour des médicaments disponibles en Europe sont situés en dehors de l'Union. ». En 1970, quelque 420 entreprises de l'industrie du médicament existaient en France. En 2017, la France ne disposait plus que de 138 sites de production de médicaments et de 92 sites de production de principes actifs ... L'Inde et la Chine possèdent chacune plusieurs milliers mes chiffres sont ceux du Pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations économiques ! La France, mais aussi l'Europe, a donc insensiblement, et pour des raisons variées- je ne néglige bien entendu pas la rentabilité -, exporté, transféré nos unités et nos savoir-faire en Asie, au détriment de notre autonomie. Plus grave, nous sommes en train de perdre notre « indépendance sanitaire » ; peut-être l'avons-nous même déjà perdue.

Il est temps pour nous, aujourd'hui, de prendre conscience que l'indépendance sanitaire est un élément essentiel de notre indépendance nationale, tout comme l'est l'indépendance énergétique. Cette remise en cause liée à la crise du covid-19 révèle le caractère gravissime de la situation. C'est pourquoi il est légitime de se pencher sur nos activités nationales en la matière et de recenser les outils dont nous disposons déjà ; c'est nécessaire si nous voulons trouver des solutions rapides, lesquelles passeront très certainement par l'Europe. Beaucoup ignorent que l'armée française joue, depuis la Révolution, un rôle en ce domaine, la pharmacie centrale des armées. Cet établissement pharmaceutique, titulaire et exploitant d'une autorisation de mise sur le marché et reconnu comme fabricant, a su préserver sa souveraineté en matière de production.

C'était au cours du second semestre 2018, voilà plus de deux ans ! Parmi les propositions les plus audacieuses que nous avions formulées figurait l'instauration d'un « programme public de production et distribution de quelques médicaments essentiels concernés par des arrêts de commercialisation, ou de médicaments régulièrement exposés à des tensions d'approvisionnement serait confié à la pharmacie centrale des armées et à l'Agence générale des équipements et produits de santé, qu'il importe de conserver. Or l'article 1 de votre proposition de loi, chers collègues du groupe communiste,

part, je suis plutôt soucieux de renforcer les outils publics tels qu'ils existent déjà. Je voterai donc contre cette proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, alors que la crise sanitaire se poursuit, que nous sommes encore dans le temps de l'action et que le rapport de la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire sera présenté demain, des premiers enseignements doivent dès à présent encore, en effet, la détresse du monde médical et la mise en danger de tous les professionnels qui ont dû poursuivre leurs activités à l'acmé de la pandémie, malgré l'impuissance du Gouvernement à les protéger.

incapables tant d'équiper les personnels travaillant en première ligne que de se procurer des masques en urgence sans dépendre des aléas et des prix du marché mondialisé. En Auvergne-Rhône-Alpes, les médicaments et les équipements de protection individuels ont longtemps manqué. l'union régionale des pharmaciens a dû, par des moyens de fortune, dépanner les pharmacies en gel hydroalcoolique dans plusieurs des départements de la région, les services déconcentrés de l'État n'ayant pas de solutions ; et c'est une association qui a assuré les livraisons.

Le système de santé français se révèle donc vulnérable aussi aux ruptures d'approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux essentiels. Ce constat ne date d'ailleurs pas de la crise du covid-19, puisque le Sénat et de très nombreux organismes alertent depuis des années sur ces ruptures d'approvisionnement.

Près d'un Français sur quatre a souffert d'une rupture d'approvisionnement. Selon la Ligue contre le cancer, 74 % des professionnels de santé ont déclaré avoir déjà été confrontés à des pénuries de médicaments

qu'il faut pouvoir produire les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la santé de leur population, s'approvisionner et les stocker de manière autonome, et cela la puissance publique qui reste le garant de cette autonomie, car la seule logique du marché ne peut y pourvoir. Nous pourrions améliorer encore la démocratie sanitaire, comme nous y encouragent les associations d'usagers du système de santé, qui demandent à être partie prenante des instances traitant du prix des médicaments et des dispositifs médicaux. Quoi qu'il en soit, entendons bien l'urgence sanitaire et les mesures qu'elle exige : la crise climatique va amplifier les crises sanitaires. Au-delà des risques pointés par les auteurs du texte, j'en appelle à notre sens collectif des responsabilités ; autrement dit, j'en appelle à- enfin ! -anticiper. En effet, si la crise du covid-19 découle indirectement de l'effondrement de la biodiversité et de la destruction des espaces naturels, d'autres facteurs, la fonte du permafrost ou les pesticides, portent en eux autant d'autres risques de maladies et de pandémies à venir. Nous devons répondre à ces enjeux par des mesures pertinentes. Dans ce contexte, la création d'un pôle public du médicament représente une première réponse, à l'échelle nationale, comme outil de régulation devant permettre d'assurer de nouveau la continuité des approvisionnements, en complément de la relocalisation des productions qui, seule, ne suffira pas. C'est pourquoi le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera cette proposition

Une enquête BVA réalisée pour France Assos Santé a montré que près d'un Français sur quatre s'était déjà vu refuser la délivrance d'un traitement pour cause de pénurie ; quatre, c'est aussi le chiffre par lequel a été multiplié le nombre annuel de signalements de tensions et de ruptures d'approvisionnement de médicaments enregistrés par l'ANSM au cours des six dernières années. Nous nous devons de remercier les professionnels de santé, prescripteurs et pharmaciens, en ville comme en établissements de santé, qui ont toujours su trouver des solutions permettant aux patients de poursuivre leur traitement. Oui, la crise sanitaire a accentué les tensions d'approvisionnement sur certains médicaments indispensables ! Je pense aux curares et aux hypnotiques, dont la consommation a augmenté de 2 000 % en l'espace de quinze jours, en pleine pandémie, au printemps. La distorsion entre l'offre et la demande, sans cesse croissante au niveau mondial, affecte l'ensemble de la chaîne du médicament. Mercredi dernier, la commission des affaires sociales a examiné le rapport de ma collègue Laurence Cohen sur la proposition de loi portant création d'un pôle public du médicament et des produits médicaux.

1 à l'article 3, crée un service public du médicament et des dispositifs médicaux. Le second chapitre crée un observatoire citoyen des dispositifs médicaux, afin de garantir la transparence des données issues de la surveillance des incidents pouvant survenir lors de l'utilisation d'un dispositif médical. Le troisième et dernier chapitre porte la taxe assise sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques de 0,17 % à 1 %, afin de mettre ces dernières à contribution pour financer ce pôle public du médicament et des dispositifs médicaux. Mes chers collègues, plusieurs dispositifs juridiques ont été élaborés pour encadrer et renforcer l'approvisionnement en médicaments. Ainsi, en 2012, puis en 2016, de nouvelles obligations incombant respectivement aux acteurs du circuit de distribution et à ceux du circuit de fabrication ont été instaurées. Force est de constater que cet arsenal juridique renforcé n'a pas permis de pallier totalement les ruptures de stock de médicaments. Aussi, en juillet 2019, Agnès Buzyn, alors ministre de la santé, avait-elle présenté une feuille de route pour lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France, dont les dispositifs sont en cours de mise en oeuvre. Cette feuille de route s'articulait autour de quatre axes promouvoir la transparence et la qualité de l'information, afin de rétablir la confiance et la fluidité entre tous les acteurs ; lutter contre les pénuries de médicaments par de nouvelles actions de prévention et de gestion sur l'ensemble du circuit du médicament renforcer la coordination nationale et la coopération européenne ; mettre en place une nouvelle gouvernance par le biais d'un comité de pilotage chargé de la stratégie de prévention et de lutte contre les pénuries de médicaments en France. pour 2020 a donné une traduction législative à certains de ces engagements. L'article 48 de ce texte crée ainsi obligation pour les industriels de constituer jusqu'à quatre mois de stocks pour tous les médicaments. Ces stocks doivent être situés sur le territoire européen et, en cas de rupture, les entreprises sont dans l'obligation d'importer à leur charge des solutions de rechange thérapeutiques pour l'ensemble des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Des sanctions financières seront appliquées si les entreprises ne constituent pas un stock de sécurité et n'informent pas l'ANSM lorsque surviennent des situations de rupture ou de risque de rupture. En outre, lors du comité stratégique de filière des industries et technologies de santé, en juin 2020, la remise du rapport Biot a été l'occasion de présenter trois axes

Dans son volet compétitivité, le plan de relance répond déjà en partie à ces défis. Il prévoit des mesures de réindustrialisation susceptibles de favoriser directement ou indirectement la relocalisation d'activités.

Vous le voyez : ici encore, le Gouvernement est à pied d'oeuvre dans nos territoires. Les pénuries de médicaments nécessitent une attention particulière des pouvoirs publics, et les mesures déjà prises sont, de ce point de vue, intéressantes ; la mise en place d'un comité de pilotage interministériel et la création d'une base de données européenne unique de mieux connaître, au niveau européen, les dispositifs médicaux mis sur le marché. À l'inverse, augmenter la fiscalité sur les entreprises pharmaceutiques au-delà de la hausse inscrite dans le PLFSS irait à l'encontre des besoins de relocalisation de ces industries et nuirait à notre compétitivité fiscale. Quant aux mesures de gouvernance visant à créer un pôle public du médicament, elles ne semblent pas adéquates, car elles risquent d'entrer en redondance avec des institutions déjà existantes comme l'ANSM et l'Inserm,

La question posée par notre proposition de loi est celle de l'accès aux médicaments. Aujourd'hui, les marchés financiers et les industriels pharmaceutiques décident des coûts des médicaments, donc de l'accès des populations Heureusement, notre pays s'est doté, en 1945, de la sécurité sociale, qui permet la prise en charge des médicaments pour les malades. Mais que se passe-t-il lorsque, comme au mois d'avril, la production des principes actifs des médicaments est interrompue ? Ni l'État ni la sécurité sociale n'ont les moyens d'agir et de produire les principes actifs à la place des laboratoires. Cette perte de maîtrise publique a tourné au casse-tête pour les patientes et les patients atteints de maladies chroniques, qui se rendent à la pharmacie la boule au ventre face aux risques de pénurie de médicaments et de rupture de soins. L'entreprise Sanofi bénéficie d'aides publiques de l'État à hauteur de 150 millions d'euros par an ; par an ; elle continue pourtant de licencier- 3 000 postes de chercheurs en moins en dix ans -et verse la moitié de ses bénéfices aux actionnaires. Oui, nous pensons que les intérêts privés sont contradictoires avec les intérêts de toutes et de tous, et qu'un pôle public de recherche et de production pharmaceutique est indispensable dans notre pays. La mainmise des laboratoires et les scandales sanitaires du Mediator et de la Dépakine ont entraîné une suspicion, parmi nos concitoyens, concernant la fiabilité des médicaments et des vaccins. La recherche effrénée des profits au détriment de la détection des effets secondaires a entamé la confiance dans les vaccins, pourtant indispensables pour se protéger, notamment, de la covid-19.

institutions telles que la pharmacie centrale des armées et la pharmacie centrale des hôpitaux de Paris. Ces deux structures publiques sont capables de produire les médicaments indispensables pour les malades hospitalisés. Il faut utiliser ces structures et les renforcer plutôt que de les affaiblir.

La concurrence effrénée entre les cliniques privées et l'hôpital public dont on réduit chaque année les moyens a fait fuir bon nombre de personnels hospitaliers. Certains services, comme en psychiatrie, se retrouvent ainsi parfois sans médecin.

La crise sanitaire de la covid-19 a mis en lumière la situation de l'hôpital public et les conditions de travail de ses personnels. Nos concitoyennes et concitoyens sont attachés à leurs hôpitaux et savent combien il est important de faire du médicament un bien commun. Ces trente dernières années ont vu l'émergence de grands progrès thérapeutiques dans la prise en charge d'un certain nombre de maladies graves. Je pense par exemple, dans le domaine des cancers, aux approches réellement innovantes, thérapies ciblées ou immunothérapies, qui ont révolutionné le pronostic de certaines affections. Ces progrès de la science et de la médecine se sont malheureusement accompagnés d'une explosion du coût de certains de ces médicaments. Il n'est désormais pas rare, pour certaines maladies, de voir des médicaments à plus de 80 000 euros par an, ce qui pose la question clé de la justification de tels niveaux de prix.

au marketing. La solution que nous proposons consiste à sortir les médicaments du marché par une réponse publique, démocratique et solidaire. Pour y parvenir, nous proposons de financer le pôle public ainsi créé par l'augmentation de la contribution des industries pharmaceutiques de 0,17 % à 1 %. Quand, en dix ans, le laboratoire Pfizer a réalisé 377 milliards d'euros de profits, une taxe de 1 % ne semble pas si excessive, d'autant que cette participation des industriels privés est un juste

nous examinons aujourd'hui une proposition de loi portant création d'un pôle public du médicament et des produits médicaux. Tout d'abord, je partage pleinement les propos de ma collègue Christine Bonfanti-Dossat, les questions qu'elle soulève comme ses conclusions. La question des ruptures de stock de médicaments est un problème récurrent depuis de trop nombreuses années ; elle touche de plus en plus de spécialités pharmaceutiques et suscite à la fois l'agacement des professionnels de santé de santé et l'incompréhension des patients, surtout ceux à qui sont prescrits des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Le Sénat, dans le cadre de sa mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins

Les causes de ces pénuries sont diverses : problèmes d'approvisionnement- une grande partie des principes actifs sont produits à l'étranger, principalement en Asie -, demande plus importante à l'échelle mondiale, problèmes sur la chaîne de fabrication, quotas imposés aux industriels, arrêt de la fabrication de médicaments matures.

en ce sens, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, un amendement visant à prendre en compte le lieu de fabrication du médicament dans le processus de fixation de son prix, et, ainsi, à favoriser les entreprises dont les usines seraient situées dans l'Union européenne, en Suisse ou au Royaume-Uni. Malheureusement, malgré la mobilisation des sénateurs et en dépit du bon sens attaché à cette mesure, l'exécutif et la majorité présidentielle n'ont pas jugé opportun de la maintenir dans le texte ; nous ne pouvons que le regretter.

Pour ces raisons, je pense qu'il serait préférable, dans un premier temps, d'optimiser la capacité de production des sites existants, la production des principes actifs, maillons essentiels de la chaîne du médicament, apparaissant bien sûr prioritaire pour retrouver une indépendance sanitaire. 2, qui porte création d'un pôle public du médicament : ce pôle se voit confier, outre une mission de production, une mission de distribution sur le territoire national. Cette mission de distribution est, à ce jour, parfaitement assurée

Leur rôle important dans la distribution de masques de l'État au début de la pandémie de covid-19 en est un exemple récent ! Ils ont parfaitement assuré cette mission. L'État a indéniablement un rôle à jouer dans la lutte contre la pénurie de médicaments. Depuis tous les gouvernements réduisent les crédits alloués au médicament sous la forme de mesures d'économies figurant dans le PLFSS. Le médicament a été, avec l'hôpital, l'une des deux variables d'ajustement des PLFSS successifs, alors qu'il ne pèse que 16,5 % du budget de la sécurité sociale.

Ainsi, depuis plus de dix ans, l'assurance maladie a mis en place des quotas. Ces quotas concernaient 400 références voilà dix ans, contre 720 références aujourd'hui ; le risque de rupture augmente de l'État, monsieur le secrétaire d'État : le cas particulier du vaccin contre la grippe. Depuis le mois de juin dernier, nous savions, vous saviez, que nous manquerions de 2 millions de doses. Preuve en est que le Gouvernement a, ces dernières semaines, acheté 2,4 millions de doses de vaccin contre la grippe. Pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas joué son rôle en anticipant cette pénurie ? Comment allez-vous vous impliquer pour que la campagne 2021-2022 se passe mieux ? Quel message allez-vous faire passer aux industriels dès ce mois de décembre, ou au plus tard au début de janvier, pour qu'on ne revive pas la même situation l'an prochain ?

Un programme public pour des médicaments qui sont en arrêt de commercialisation paraît facile à envisager. En revanche, comment aborder la question pour les médicaments qui sont en rupture d'approvisionnement ? Comment anticiper ces ruptures ? Certes, les laboratoires ont l'obligation légale de déclarer les risques de rupture, mais comment un pôle public du médicament pourrait-il avoir la réactivité suffisante pour corriger ces risques ? Comment prendrait-il concrètement la main ?

L'examen de cette proposition de loi ne se réduit pas à un affrontement entre deux visions antagonistes de la politique du médicament : l'une du tout-État et de la planification vertueuse contre l'autre du tout libéral, qui laisserait un boulevard aux laboratoires et à leurs intérêts de court terme. À titre personnel, je considère que l'équilibre se situe à la frontière entre ces deux sphères. La concurrence est vertueuse dans le sens où elle est source d'innovation et de progrès continu. Toutefois, l'État a effectivement un rôle de régulateur à jouer, en particulier sur un sujet qui concerne la santé de nos concitoyens.

Monsieur le ministre,

-, a décidé d'arrêter la commercialisation d'Immucyst, un vaccin BCG utilisé comme antinéoplasique, privant ainsi de nombreux patients d'un traitement qui leur aurait permis d'éviter une ablation de la vessie. Quels outils avons-nous pour contraindre ce laboratoire à

pense, par exemple, à l'accueil de patients français par les hôpitaux allemands, mais aussi à l'envoi de médecins cubains en Italie. Le Président de la République a indiqué lors du dernier sommet du G20 que le vaccin contre la covid-19 devait être considéré comme un « bien public mondial » et être vendu à prix coûtant. Bien évidemment, nous partageons cette position, d'autant que la pandémie a tué des millions de personnes dans le monde. Il faut donc une solidarité

ces derniers mois. Le renoncement aux soins, mais aussi les errements de communication sur la recherche et la stratégie médicamenteuse pour enrayer cette épidémie en sont les stigmates. Cette tendance, c'est le recul de la place accordée aux usagers de santé et à leurs représentants.

Le rôle de cette nouvelle entité serait de garantir une meilleure transparence des données issues de la surveillance des incidents pouvant survenir lors de l'utilisation d'un dispositif médical, par exemple. Cet observatoire citoyen appelle, par son intitulé, à accorder enfin à l'usager la place qui lui est due, car nous le savons tous : l'opacité fait naître la défiance.

sont prêts. Si un enseignement doit être tiré de cette crise sanitaire, c'est bien qu'il est nécessaire de réinstaurer au sein du système de santé et des entités qui le composent plus de démocratie sanitaire.

ou en voie de l'être dans le cadre de la politique d'ouverture de l'ANSM. Plusieurs éléments concourent ainsi, ou concourront bientôt, à cette transparence que, comme nous, vous appelez de vos voeux : d'une part, le rapport d'activité de l'ANSM, qui comporte chaque année une synthèse des données de vigilance et les faits marquants de l'année

aujourd'hui pour les données de pharmacovigilance. En outre, il convient de rappeler que, depuis le mois de juillet 2019, dans l'ensemble des instances d'expertise scientifique de l'Agence siègent des représentants des patients et des représentants d'usagers du système de santé.

des associations de patients, deux titulaires et deux suppléants. De plus en plus, l'ANSM procède à des consultations et à des auditions publiques des parties prenantes, lesquelles font l'objet d'une diffusion en direct sur internet, de même que les ordres du jour et les comptes rendus de ces séances. Il ne nous semble donc pas nécessaire de créer par voie législative une instance supplémentaire,

mais la pandémie et la manière dont nous traitons la question du vaccin démontrent qu'il faut changer de logique et ne plus laisser la main aux groupes industriels actuels. Souvenons-nous de la déclaration du directeur France de Sanofi,

sinon nous nous préparons des catastrophes sanitaires sur l'autel des rendements des groupes pharmaceutiques.

pourtant bien parce qu'elle existe que nous pouvons interpeller le Gouvernement et lui demander pourquoi cette instance de démocratie sanitaire n'a jamais été consultée. Ce qui existe à l'ANSM sur le médicament

en termes de démocratie sanitaire sur la question du médicament. C'est pour cela que nous avons soutenu cette disposition et que nous regrettons que le Sénat ne fasse pas ce petit pas en avant sur cette question. La parole est à M.

Les ruptures ou pénuries recensées sont passées de 44 en 2008 à plus de 1 200 en 2019, soit 30 fois plus Aucune classe thérapeutique n'est réellement épargnée. Les pénuries et ruptures touchent des catégories variées de médicaments et de produits de santé : des antibiotiques aux traitements utilisés contre le VIH, les cancers, les vaccins ou encore les médicaments utilisés dans les protocoles de fin de vie. Les médicaments et produits de santé sont soumis aux logiques de l'offre et de la demande et des profits. Les industriels peuvent donc négliger des marchés qui ne leur semblent pas rentables, même lorsqu'il s'agit de molécules indispensables. De plus, pour réduire les coûts de main-d'oeuvre, les groupes ont délocalisé leur production. Nous dépendons désormais à 80 % de la Chine et de l'Inde. le Gouvernement a de son côté refusé de réquisitionner les sites de production récemment fermés, qui disposaient pourtant de toutes les infrastructures pour produire ces médicaments, comme le site de Sanofi à Romainville et celui de Famar à Lyon.

qui confondent les missions du public avec celles du privé. Le public ne cherche ni la rentabilité ni le profit : il sert l'intérêt commun.

Les articles de la proposition de loi ayant été successivement rejetés par le Sénat, je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a plus de texte. En conséquence, la proposition de loi n'est pas adoptée. La parole est à Mme

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous abordons un thème cher au sénat, celui de l'aménagement numérique du territoire. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'une question essentielle pour nos concitoyens, comme l'a démontré avec acuité la crise de la covid-19. Cette crise a révélé de nouvelles fractures au sein de notre société : aux fractures sociales

acuité la crise de la covid-19. Cette crise a révélé de nouvelles fractures au sein de notre société : aux fractures sociales entre les premiers de cordée et les premiers de corvée se sont ajoutées des fractures territoriales et numériques dans l'accès aux services publics. Ainsi, la question de l'accès à une connexion internet de qualité comme au réseau téléphonique mobile a été cruciale pour nombre de nos concitoyens dans leur rapport au monde durant le confinement. Grâce à une bonne connectivité, certains ont pu profiter de leurs proches, mais également poursuivre leur travail à distance, suivre des cours, des formations, accéder aux collections des musées, à la culture en ligne et aux divertissements, ou encore régler des problèmes administratifs, inscrire leurs enfants aux activités, payer la cantine, faire leurs courses livrables à domicile ... Bref, ils ont pu continuer de vivre dans les conditions permises par l'État d'urgence sanitaire. Pour d'autres, l'isolement physique a été conjugué à un isolement numérique, une telle situation étant insupportable moralement, mais également particulièrement handicapante. De ce constat, nous tirons une leçon. Les réseaux de télécommunications sont à l'image des réseaux de communications au XIX siècle : un levier puissant d'aménagement du territoire et de désenclavement, un outil d'intégration au monde.

Faute d'une telle spécification, corollaire d'un nouveau droit au numérique qui reste à conquérir, la place laissée à l'initiative privée a été prépondérante. L'urgence à l'époque a été de démanteler le monopole d'alors, celui de France Télécom, devenu Orange, pour permettre, au nom des directives européennes et de la concurrence, à d'autres opérateurs de s'installer. Une telle situation devait être favorable aux usagers, devenus des clients. Or que constate-t-on ? Ce changement de paradigme et la succession des différents plans n'ont pas permis d'avancer vers une couverture intégrale des territoires, et trop de nos concitoyens restent toujours sur le bord des routes numériques. Alors que le plan France Très haut débit, adopté le 28 février 2013 par le Gouvernement, a fixé l'objectif d'une couverture intégrale du territoire en très haut débit d'abord en 2022, puis en 2025, nous en sommes malheureusement encore loin. Avec ce plan, 80 % de la population devrait être directement reliée à la fibre optique. Ce plan très haut débit prévoit de mobiliser les acteurs privés et publics, pour un investissement total évalué à 20 milliards d'euros. Pour ce faire, le territoire est coupé en deux. Sur le territoire le plus dense, représentant 57 % de la population, les opérateurs s'engagent à déployer des réseaux de fibre privés mutualisés de très haut débit dans le cadre de conventions signées avec l'État et les collectivités concernées. Le déploiement des réseaux privés nécessite un investissement des opérateurs de 6 milliards à 7 milliards d'euros. Pour le reste du territoire, qui représente 43 % de la population, mais 90 % du territoire,

Ceux-ci sont aujourd'hui frappés d'une faiblesse qui tient à la difficulté, une fois même le réseau créé, de trouver des opérateurs pour s'y inscrire. Ainsi, dans les RIP, seuls 26 % des prises installées bénéficient de l'offre de plus d'un opérateur. Par ce découpage, le plan entérine et poursuit un schéma bien connu, dans lequel on privatise les profits et socialise les pertes. Là où la rentabilité est assurée, les opérateurs interviennent et, là où ce n'est pas le cas, la puissance publique se substitue

Dans les zones intermédiaires, pas tout à fait denses, mais suffisamment pour se passer de l'initiative publique, on a recours aux appels à manifestation d'intérêt, laissant encore le secteur privé répondre à des questions relevant de l'intérêt général. général. Le déploiement de réseaux publics par les collectivités territoriales représente un investissement de 13 milliards à 14 milliards d'euros. Les recettes d'exploitation et le cofinancement des opérateurs privés doivent financer la moitié de cet investissement, limitant le besoin de subventions publiques à 6,5 milliards d'euros. Sur cette somme, le plan France Très haut débit prévoit un double soutien financier pour les projets des collectivités d'une part, une subvention de l'État de 3,3 milliards d'euros et, d'autre part, l'accès à des prêts à des taux préférentiels. En décembre 2017, le Gouvernement a pourtant stoppé les subventions et fermé le guichet chargé de distribuer ces aides aux collectivités. suite d'une forte mobilisation des territoires, le guichet a rouvert en décembre 2019, avec un financement limité à 140 millions d'euros. Dans la loi de finances pour 2020, ces sommes sont même passées à 440 millions d'euros. Le Sénat a obtenu, dans la troisième loi de finances rectificative, une rallonge de 30 millions d'euros. Le plan de relance, dans le cadre de la loi de finances pour 2021, prévoit, lui, de nouvelles autorisations d'engagement, à hauteur de 240 millions d'euros. Autrement dit, en cumulé,

Par ailleurs, dans un rapport du 31 janvier 2017, la Cour des comptes a estimé que le projet devrait dépasser la durée et le budget initiaux, pour passer de 20 milliards à 35 milliards d'euros et s'étaler jusqu'en 2030, ce qui soulève de nouvelles questions de financement. financement. Ces chiffres étant très décevants- aujourd'hui seuls un peu plus de 50 % des locaux disposent d'une couverture en très haut débit -, nous considérons qu'il convient de changer de modèle. L'effort public doit être réévalué de manière globale, afin de redonner un cadre à l'investissement et à l'action publique en faveur de l'aménagement numérique des territoires. L'intervention publique de l'État ne peut se limiter à une politique de guichet ou à des appels à manifestation d'intérêt, encore moins à des enchères publiques, comme avec la 5G, qui pose pourtant tant de problèmes éthiques et politiques, comme l'a souligné la Convention citoyenne sur le climat. L'intervention privée doit donc être mieux encadrée.

pour un réseau filaire ou de 3 % du chiffre d'affaires. Pour autant, force est de reconnaître que ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune mise en oeuvre, alors même que, à la fin du premier trimestre 2020, Orange et SFR n'avaient rendu raccordables respectivement que 67 % et 75 % des sites d'investissement). Je crains donc que ces mesures ne soient assez peu dissuasives. La question des modalités de construction et de gestion des infrastructures numériques reste entière. Elle est prioritaire. Pourquoi permettre aux opérateurs privés d'être propriétaires des infrastructures dans les zones denses et rentables et les exonérer de cette obligation dans les zones non rentables ? Pourquoi ne pas avoir soit séparé partout les infrastructures et les activités d'opérateurs, à l'image par exemple du rail, soit conservé un modèle unifié qui aurait permis de basculer, grâce à la rente du cuivre, au fibrage de l'ensemble des territoires ? Nous sommes aujourd'hui dans un modèle hybride, inopérant pour remplir ses missions d'intérêt général. Nous considérons ainsi qu'il est nécessaire de créer un opérateur national, propriétaire des réseaux, et dont le financement serait assuré à la fois par les opérateurs et par l'État. Il s'agit de doter cet opérateur de ressources mutualisées, pourquoi pas au travers d'un fonds dédié, alimenté par les entreprises sur leurs bénéfices, souvent considérables et si souvent décriés comme le résultat d'ententes. Les actions de SFR, Bouygues et Orange se portent toutes très bien, leurs résultats étant positifs, même avec la crise ! Dans le modèle que nous vous proposons, toutes les recettes de l'opérateur de réseau seraient obligatoirement réinvesties dans le développement et l'entretien du réseau existant. Il s'agirait ainsi de permettre la mutualisation des recettes des zones denses pour couvrir les besoins des zones moins denses, ce qui serait une avancée considérable. Rappelons pour finir que la Commission européenne a fixé pour 2025 l'objectif d'une couverture totale des locaux à 100 mégabits par seconde, soit la mise en place de la fibre jusqu'à l'ensemble des abonnés. La France se doit donc de créer les moyens d'atteindre ces objectifs afin d'éviter d'aggraver des fractures territoriales en créant de nouveaux déserts numériques,

Nous voulons montrer, à travers cet exemple, combien des territoires entiers de notre pays ont été oubliés du fait d'un désengagement de l'État, et ce depuis plusieurs années. Encore très récemment, la mise aux enchères des fréquences de la 5G a été une belle illustration de ce laisser-faire coupable. L'attribution de ces fréquences, qui s'est faite au plus offrant et a rapporté 2,7 milliards d'euros, n'avait pour seul but que de faire entrer de l'argent frais dans les caisses de l'État. Avouez, mes chers collègues, que c'est curieux en termes de politique publique, d'autant que les opérateurs eux-mêmes avaient alerté le Gouvernement sur le caractère non urgent de ces enchères au regard des retards existants concernant la 4G. Cette démarche est d'autant plus curieuse que le passage à la 5G devrait également priver d'accès près de 4 000 foyers dans quarante départements particulièrement enclavés. Ce nouvel épisode confirme ainsi les schémas existants d'intervention publique et privée structurés autour d'une socialisation des pertes et d'une privatisation des profits. Au-delà du modèle économique, ces éléments nous interrogent également en matière de stratégie industrielle nationale et de démocratie. Je prendrai encore une fois l'exemple de la 5G. Cette technologie, par ses performances en termes de connectivité, est une innovation d'importance.

les questions qui se posent aujourd'hui concernant son développement ne relèvent pas de ces enjeux industriels ou d'aménagement ; le seul prisme est celui de la rentabilité. Nous allons donc continuer de multiplier les infrastructures et les pylônes en zone dense

Car, mes chers collègues, c'est aussi une question démocratique ! Il apparaît nécessaire que le Parlement se dote enfin réellement d'un plan stratégique de développement numérique adossé à la création d'un véritable service public permettant de garantir le droit le droit au très haut débit pour tous. Ce plan doit être présenté et voté au Parlement. Il devrait fixer des objectifs non seulement de connectivité et de couverture du territoire, mais également industriels, liés au développement de ces technologies, adossés à des outils publics et à des études fiables, ce qui manque aujourd'hui et nourrit toutes les défiances. Il nous faut reconstruire un pôle public des télécommunications responsable de ce service public. La privatisation de France Télécom a été une folie économique et sociale. Alors que la rente du cuivre aurait permis de financer la fibre sur tout le territoire, l'État a préféré brader ce fleuron industriel. Or nous avons besoin d'une stratégie industrielle nationale dans le secteur du numérique, c'est une évidence. Les enjeux sociaux sont aussi importants un renforcement de la prise en charge de l'accès des plus fragiles, car il s'agit bien d'un service essentiel, nous l'avons vu durant le confinement. Enfin, un tel plan doit fixer des objectifs environnementaux de sobriété. Cette exigence, qui s'exprime de plus en plus fortement, doit être prise en compte. Pourtant, aujourd'hui, le développement numérique reste un angle mort démocratique, le Parlement étant simplement appelé à constater ou non le respect par les opérateurs privés de leurs engagements peu contraignants dans le cadre du plan France Très haut débit et du contrôle de l'Arcep. De même, alors que les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont exigé un moratoire sur le développement de ces technologies, l'exécutif leur a répondu par le dédain en les qualifiant d'« traduisant un mépris tout jupitérien. Nous pensons que l'utilité publique de ces usages justifie des débats avec la Convention citoyenne, mais aussi avec les associations, les élus et le Parlement. Tels sont, mes chers collègues, les éléments que je souhaitais vous soumettre, en complément de la présentation de notre proposition

car j'en partage le constat, à savoir celui d'une fracture numérique persistante au sein de notre société. La crise sanitaire a mis en lumière le caractère essentiel des réseaux numériques pour la continuité des activités de la Nation, qu'il s'agisse de continuer à apprendre, à travailler, à se soigner la téléconsultation, ou simplement de garder un contact avec nos proches. Relever ce défi nous permettra collectivement de désenclaver nos territoires et de les rendre plus attractifs pour les entreprises et nos concitoyens. Pour toutes ces raisons, je partage le constat de nos collègues du groupe CRCE.

Force est de rappeler que le service universel découlant de la directive européenne portant création du code européen des communications électroniques intègre l'accès au haut débit et non au très haut débit. Il est vrai qu'un doute existe sur la possibilité d'atteindre en 2020

Ce doute, mes chers collègues, semble bel et bien confirmé sachant que le guichet Cohésion numérique des territoires, qui permet, dans l'attente de l'arrivée de la fibre, de financer des équipements pour une connexion non filaire, est trop peu utilisé. Seuls 600 000 euros ont été décaissés au 30 juin Nous sommes donc très loin des 100 millions d'euros budgétés. Toutefois, et j'y reviendrai, les financements sont maintenant sur la table et les rythmes de déploiement sont globalement satisfaisants en matière de très haut débit. les auteurs de la proposition de résolution considèrent qu'il convient de s'interroger sur l'opportunité de créer un véritable pôle public des télécommunications afin de garantir le service universel et la maîtrise publique des infrastructures numériques. que la planification et l'initiative publique valent déjà dans les zones rurales et peu denses, où a été reconnue, au début des années 2010, la carence de l'initiative privée. Ainsi, dans ces territoires, le déploiement s'opère sous l'autorité des collectivités territoriales, avec un soutien financier de l'État, des réseaux d'initiative publique. Ailleurs, en revanche, la logique de planification n'a pas été retenue, car il a été jugé préférable de s'appuyer sur une logique concurrentielle, considérant que le marché pouvait aboutir à un déploiement dynamique. Cela n'empêche pas, dans cette zone d'initiative privée, la souscription d'engagements contraignants, afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs par les acteurs privés : c'est la logique des fameuses zones AMII. Dès lors, la logique de planification de la présente proposition de résolution n'est ni celle du plan France Très haut débit ni celle du Sénat, et je considère qu'il convient de laisser fonctionner la logique concurrentielle, qui aboutit à des rythmes de déploiement satisfaisants, voire inédits, avec par exemple l'installation de près de 5 millions de prises en 2019 pour la fibre optique jusqu'au domicile. Dès lors, la logique hybride actuelle semble pertinente, à condition que le régulateur puisse sanctionner la non-atteinte des objectifs, j'y reviendrai également. fibre optique. Ils estiment nécessaire de revoir les architectures de financement des réseaux d'initiative publique afin que l'État accorde un soutien exceptionnel aux collectivités volontaires, Il est vrai que, en 2019, vingt-cinq départements n'avaient pas encore finalisé leur plan de financement pour la généralisation de la fibre optique, illustration de crédits insuffisamment déployés par l'État dans ces territoires. Le Sénat, ainsi que la commission que je préside, avait régulièrement alerté le Gouvernement sur ce sujet. Après une première rallonge de 30 millions d'euros, sur l'initiative du Sénat, dans la troisième loi de finances rectificative, le plan de relance nous apporte enfin satisfaction. Celui-ci prévoit en effet de nouvelles autorisations d'engagement à hauteur de 240 millions d'euros, offrant de la visibilité pour la généralisation de la fibre d'ici à 2025. Il s'agit d'une victoire politique majeure pour notre assemblée et notre commission, engagées dans ce combat pour assurer la couverture numérique des territoires. À cet égard, je tiens à saluer nos collègues Hervé Maurey et Patrick Chaize, qui se sont particulièrement investis sur ce sujet. de ce texte souhaitent des mesures plus contraignantes afin que les opérateurs privés respectent les obligations qu'ils ont contractées. La couverture intégrale des zones AMII accuse en effet un certain retard pour lequel la crise sanitaire ne constitue pas une explication suffisante. À la fin du premier trimestre 2020, Orange et SFR avaient rendu respectivement 67 % et 75 % des sites en zones AMII raccordables, ce qui est assez loin de l'objectif souscrit auprès de l'Arcep.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera contre cette proposition de résolution. La parole

Un État moderne est un État qui sait donner des impulsions sans se substituer aux acteurs de la société- citoyens, associations, entreprises, collectivités territoriales l'État épaule leurs efforts, en leur donnant les moyens d'agir par eux-mêmes. » Ces paroles, prononcées le 26 août 1999 par Lionel Jospin, alors Premier ministre, lors de l'Université d'été de la communication à Hourtin, définissaient à l'époque la stratégie du Gouvernement pour la société de l'information. Il était temps d'agir, car si la France avait réussi son plan téléphone en 1970, ouvrant dix ans plus tard la voie au célèbre et populaire Minitel, elle avait raté le plan câble les années suivantes et commençait à accumuler du retard dans ce que l'on appelait à l'époque les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais il faudra tout de même attendre février 2013 pour que les fondamentaux de cette stratégie soient posés, sous l'impulsion de François Hollande, avec le plan France Très haut débit. Celui-ci reposait sur un constat simple : la couverture intégrale et rapide du territoire représente des investissements tels qu'ils nécessitent bel et bien un partage des rôles entre initiative publique et privée. Dans les zones très denses, soit 57 % de la population, l'initiative privée doit se mobiliser et, dans les zones moins denses, après appel à manifestation d'intention d'investissement, là où il y a donc une carence constatée du privé, c'est à la puissance publique d'agir par le biais des collectivités, et c'est à l'État de les accompagner, à l'aide d'un guichet de financement doté initialement de 3,3 milliards d'euros. Il est à noter que les collectivités ont la possibilité de se refinancer en percevant des redevances d'utilisation. La question que nous devons nous poser est de savoir si ce modèle est efficient. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il va permettre d'atteindre les objectifs de la couverture intégrale, soit plus de 40 millions de logements et de locaux à raccorder d'ici à 2025. Nous pouvons constater que le rythme des déploiements est soutenu, de l'ordre de 4,8 millions de prises en 2019 ; quasiment le même nombre est attendu en 2020, malgré la crise sanitaire. Les acteurs privés du secteur investissent de l'ordre de 10 milliards d'euros par an, soit plus de 50 milliards d'euros depuis six ans. Concernant les zones moins denses, nous partageons l'idée que l'État doit, plus que jamais, continuer d'apporter son soutien financier aux réseaux d'initiative publique portés par les collectivités, afin de sécuriser le déploiement de la fibre dans les territoires isolés ou encore mal desservis. Comme l'a souligné Jean-François Longeot, notre assemblée a pesé de tout son poids et les crédits complémentaires disponibles s'élèveront à 550 millions d'euros, dont 240 millions issus du plan de relance, ce qui offre enfin une visibilité aux vingt et un départements n'ayant pas complété à ce jour leur plan de financement. Certes, quelques incertitudes demeurent sur le futur cahier des charges, sur les raccordements complexes, mais l'horizon semble dégagé. Une des particularités du plan de 2013 est d'avoir renforcé l'action du régulateur.

À ce titre, le traitement des 43 retards au regard des 445 premiers sites du de la couverture ciblée sera un véritable test. L'Arcep a toujours su faire preuve de fermeté, si bien que les relations ont parfois été tendues avec les opérateurs. Citons, pour mémoire, la question prioritaire de constitutionnalité, qui démontre, à juste titre, qu'une réflexion sur un éventuel renforcement de ses pouvoirs peut être engagée, notamment sur les impacts environnementaux des réseaux, tout en veillant bien évidemment à l'équilibre des relations entre les acteurs. De même, l'Arcep devra s'approprier de nouveaux sujets. Ainsi, dans les zones très denses où les déploiements sont sous la totale responsabilité de l'initiative privée, on constate des retards c'est notamment le cas à Bobigny, à Lille et à Clermont-Ferrand. Ces retards sont-ils fortuits ou dus aux stratégies commerciales de certains opérateurs, qui ne veulent pas se départir d'abonnements souscrits en ADSL ? L'Autorité devra y répondre.

au risque de troubler mes collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, je vais être assez bienveillant avec les dispositions de cette proposition de résolution. D'abord, je souscris aux considérants : comment pourrait-il en être autrement ? Surtout, je peux faire mien le raisonnement qui les a conduits à formuler chacune de leurs quatre propositions. Cependant, pour ne pas ébranler davantage les auteurs de la présente proposition de résolution, je préfère immédiatement les prévenir que je voterai contre ce texte.

Je n'ai pas d'idéologique sur la propriété publique des réseaux de télécommunications : les réseaux d'initiative publique (RIP) en sont une forme décentralisée. Et c'est précisément

secrétaire d'État, mes chers collègues, hasard du calendrier, hier, Paul-Henry Martin, habitant Pierre-Châtel dans le sud de l'Isère, m'interpellait pour me signaler les difficultés que rencontre sa commune pour être raccordée à la fibre optique. La semaine dernière, un maire de ma région, le Trièves, m'indiquait qu'un jeune couple avait renoncé à s'installer dans sa commune, faute de liaisons internet et mobile. Voilà quelque temps, un artisan me racontait qu'il était obligé de prendre sa voiture pour télécharger un dossier d'appel d'offres depuis un village mieux desservi. Je pourrais vous donner bien d'autres exemples, monsieur le secrétaire d'État. C'est- hélas ! -le quotidien de nombreux habitants en zones rurales, et plus encore en montagne. Selon les données de l'Arcep du mois de juillet 2020, près d'un tiers des foyers français n'ont toujours pas accès à la fibre. Son déploiement est devenu un enjeu de politique locale ; la réalisation est assurée en grande partie par les départements. Or, force est de le constater, malgré les millions d'euros de fonds publics européens, régionaux, intercommunaux et même communaux

un modèle basé sur la rentabilité et la concurrence au détriment du service rendu aux habitants. Corriger ce modèle défaillant, c'est tout l'objet de la présente proposition de résolution, que j'ai l'honneur d'avoir cosignée avec la présidente Éliane Assassi. Je remercie d'ailleurs vivement nos collègues du groupe CRCE d'avoir inscrit ce texte à l'ordre du jour L'État doit redevenir moteur en matière d'aménagement du territoire. Comme d'habitude, les opérateurs privés s'intéressent seulement aux zones denses qui leur assurent un retour sur investissement. On ne peut nullement compter sur eux pour équiper les 43 % d'habitants des zones peu denses et non conditionnées. Comme pour le rail, on aurait pu imaginer, même si ce n'est pas la panacée, un modèle où l'État déploie les réseaux, en détient la propriété et les loue aux opérateurs privés. Sans cohérence et sans faire d'économie, on a laissé les opérateurs déployer les réseaux, souvent sans concertation et sans assurer la couverture totale du territoire. Pis, pour le déploiement de l'internet mobile, on a laissé les trois grands opérateurs installer chacun leurs propres antennes relais, sans incitation à la mutualisation, multipliant ainsi inutilement les infrastructures. Quelle aberration écologique ! Quel gâchis économique ! Et je ne parle même pas du déni démocratique puisque les habitants ne sont même plus informés en amont de l'installation de ces antennes de stabiliser ce système hybride et bancal, l'État et les collectivités doivent investir des milliards d'euros pour se substituer aux opérateurs privés et compléter la couverture du pays. C'est l'objet du plan France Très haut débit, lancé en 2013. On mesure vingt ans plus tard toute la vision politique des gouvernements qui ont privatisé France Télécom ! Faute d'opérateur national, d'une stratégie nationale cohérente et d'une expertise publique suffisante, voilà la France incapable de fibrer correctement son petit territoire en moins d'une décennie. Monsieur le secrétaire d'État, la promesse présidentielle de parvenir à la fin de l'année 2020 au 100 % de haut et très haut débit n'a pas connu plus de succès que celle de sortir du glyphosate à la même échéance. du plan France Très haut débit ont déjà été repoussés à 2025. Pour tenir cet horizon lointain, que nous impose d'ailleurs la Commission européenne, l'État doit accompagner les collectivités locales. Il est nécessaire, comme le proposent les auteurs de la résolution, de revoir l'architecture de financement des réseaux d'initiative publique et d'accorder un soutien exceptionnel aux collectivités les plus en retard. Faute de soutien financier de l'État, de sanction effective et de mesures plus contraignantes à destination des opérateurs, nombre de nos concitoyens continueront à vivre des années durant en zone blanche. Monsieur le secrétaire d'État, pour le seul intérêt de quelques entreprises, le gouvernement auquel vous appartenez ne pense qu'à déployer en urgence la 5G dans les grandes villes, sans débat démocratique et sans attendre le résultat des études sanitaires. Vous invoquez les besoins de téléconsultations de médecine en zone rurale dans des endroits où l'on ne peut parfois même pas envoyer un mail ou passer un coup de téléphone. Loin de résorber la fracture numérique et la fracture territoriale, votre politique l'aggrave. Vous pourriez conditionner le déploiement de la 5G à la complétude préalable du réseau fibre ou 3G.

que le vote du Sénat ne soit pas unanime. La Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le numérique est plus que jamais essentiel dans nos vies, aussi bien pour apprendre, pour travailler, pour avoir accès à ses droits, pour se divertir que pour consommer. Le confinement et les contraintes sanitaires ne font qu'accentuer ce constat. Le numérique n'est pas un luxe. C'est un droit essentiel au fonctionnement de notre pays. En effet, il faut garantir à chaque citoyen, en ville comme à la campagne, en métropole comme outre-mer, un accès à internet performant avec la construction ou le déploiement d'équipements de qualité. En France, le déploiement du numérique et du mobile est bien en cours et s'accélère. L'infrastructure numérique est un bien de première nécessité. C'est pourquoi le Gouvernement en a fait un marqueur de son action. C'est également un élément clé de la cohésion des territoires, d'inclusion des citoyens et de compétitivité de notre économie.

effet, au mois de janvier 2018, le Gouvernement a conclu un accord historique avec les quatre opérateurs de téléphonie mobile pour généraliser la 4G en France. Pour ces opérateurs, cela représente cinq engagements forts et contraignants convertir les pylônes 2G et 3G existants en pylônes 4G ; assurer la couverture mobile dans des zones stratégiques non ou mal couvertes ; généraliser la 4G dans les transports, dont 55 000 kilomètres d'axes routiers et 23 000 kilomètres de voies ferrées ; optimiser le passage de la 4G à l'intérieur des bâtiments

Ce contrôle est totalement transparent puisque les indicateurs de suivi de mise en oeuvre des engagements sont accessibles sur le site internet de l'Autorité. De plus, dans la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, le et du numérique, le Gouvernement a donné des moyens complémentaires pour atteindre ces objectifs ambitieux de couverture de l'ensemble du territoire en très haut débit. Il est d'ailleurs à noter que le Sénat a fortement contribué à enrichir le texte lors de son examen. Il faut aussi mettre l'accent sur l'évolution déterminante que constituent pour la ruralité la couverture en très haut débit et la résorption des zones blanches de téléphonie mobile. En effet, quand le très haut débit et la téléphonie mobile 4G, puis la 5G 5G innerveront le monde rural, un obstacle majeur à l'installation d'entreprises et à l'arrivée de travailleurs qualifiés indépendants sera levé, répondant ainsi aux préoccupations de M. Gontard. C'est tout à fait essentiel, structurant. Cela induit une nouvelle forme d'aménagement du territoire et de nouveaux modes de vie pour les Français. L'État a engagé un plan France Très haut débit. En 2022, 100 % des Français seront éligibles au très haut débit, dont 80 % grâce à la fibre optique. Le Gouvernement veut aller plus loin et se fixe un objectif ambitieux : la généralisation de la fibre optique jusqu'à l'abonné sur l'ensemble du territoire à l'horizon 2025. Dans le cadre du plan France Très haut débit, 75 % des départements ont déjà prévu la généralisation de la fibre optique sur leur territoire d'ici à 2025. Si les départements sont généralement les maîtres d'ouvrage, l'État est le principal financeur, avec un apport historique de 3,3 milliards d'euros sous ce quinquennat, abondé par des crédits européens. Le plan de relance permet d'ajouter 240 millions d'euros au bénéfice de cette priorité politique pour en accélérer encore la mise en oeuvre. Un investissement de cette ampleur est inédit et permet d'accélérer la couverture numérique du territoire. D'ici à la fin de l'année, quasiment tous les Français auront un accès à internet haut débit. Le très haut débit, lui, sera accessible d'ici à 2022. L'accès à internet par la fibre optique sera généralisé à l'horizon 2025. Ces trajectoires et les moyens dévolus pour les atteindre font de ce quinquennat le plus volontariste pour renforcer la couverture du territoire depuis des décennies. En zone d'initiative publique- cela concerne en premier lieu les territoires ruraux -, au deuxième trimestre de 2020, ce sont 4,3 millions de locaux qui ont été raccordés au réseau fibre à l'abonné, contre 2,5 millions à la fin du deuxième trimestre de 2019, soit une hausse de 72 % en un an. Le Gouvernement a ensuite pour objectif la généralisation de la 4G sur l'ensemble du territoire national. À ce jour, 76 % du territoire est couvert par tous les opérateurs, contre 45 % seulement au 1 janvier 2018. Un effort important a également été fourni pour améliorer la couverture mobile dans les zones blanches ou mal couvertes. Alors qu'au cours des quinze dernières années, seulement 600 nouveaux pylônes avaient été inaugurés, ce sont plus de 2 000 nouveaux pylônes qui vont être déployés en deux ans. Parmi ceux-ci, 462 ont déjà été mis en service, et le rythme des inaugurations est soutenu. Le très haut débit devrait également nous permettre d'avancer sur un sujet stratégique pour la population française, particulièrement en zone rurale : la prise en charge sanitaire de la population, avec la télémédecine, qui continue de se développer puisque nous sommes passés de 50 000 consultations l'année dernière à un million au cours du premier confinement.

Dans les deux cas, la crise que nous vivons depuis plusieurs mois a fait émerger de manière encore plus prégnante le besoin de réformes et d'accélération de celles qui sont déjà engagées. Sur le constat, nous ne pouvons qu'adhérer à cette proposition de résolution. Le numérique renforce l'accès de nos concitoyens aux services, à plus forte raison en période de confinement, de distanciation physique et de gestes barrières : démarches administratives, télémédecine, accès à l'information, aux savoirs et à la culture, ouverture sur le monde et, bien sûr, télétravail, dont la montée en puissance au printemps a été brutale, nous invitant à accélérer le déploiement du très haut débit. Le numérique est également un outil de désenclavement et d'attractivité des territoires, en particulier en zone rurale, où l'accès aux services est plus difficile. La polarisation de notre modèle d'aménagement du territoire autour des métropoles a entraîné pour de nombreuses régions une perte de population avec, en corollaire, une inquiétante diminution de l'accès aux services essentiels. Or, si l'on veut désengorger les métropoles et relancer la dynamique des zones rurales et périurbaines, il faut nécessairement un accès internet de qualité partout et pour tous. On ne peut nier le besoin exprimé depuis le début de la crise sanitaire par de nombreux Français, qui aspirent à une vie hors des centres-villes. À nous de leur proposer des solutions pour qu'ils réalisent leur rêve et celui de tous les élus des territoires que nous représentons.

Après des investissements jugés insuffisants, l'État a inscrit dans le projet de loi de finances rectificative et dans le plan de relance des crédits supplémentaires, le total s'élevant à 550 millions d'euros. Selon l'Arcep, plus 10 millions de locaux seront abonnés à la fibre à la fin de l'année, soit 50 % de plus qu'en 2019. À ce rythme, l'ensemble des 41 millions de locaux français pourraient être fibrés d'ici à fibrés d'ici à quatre ans. L'Arcep indique que 96 % du territoire est couvert par la 4G par au moins un opérateur. Les chiffres sont donc encourageants.

régie Auvergne Numérique permettra bientôt à 91 % des locaux auvergnats d'être couverts par la fibre, grâce aux 300 millions d'euros investis par la région, les quatre départements, l'État et l'Europe. Nous pensons qu'il faut accompagner les initiatives déjà engagées plutôt que de renverser cet équilibre fragile. Les budgets alloués par l'État et l'aide que l'ANCT apporte aux collectivités devraient permettre d'accélérer le déploiement du très haut débit dans les zones qui en sont encore exclues. est le sujet qui nous préoccupe : seul un quart des Français sont raccordables à la fibre en zone rurale, contre 80 % dans les grandes villes. Pour cela, cette proposition de résolution appelle à la création d'un nouveau droit, sous la forme d'un service universel. C'est ce que prévoit déjà le plan France Très haut débit à l'horizon 2025 ... Cet horizon peut, en effet, paraître bien lointain pour ceux dont la connexion défaillante renforce les fractures territoriales que nous ne parvenons déjà pas à résorber. Nous sommes toutefois convaincus qu'une nouvelle réforme n'est pas la bienvenue en la matière. C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra sur ce texte. Il faut avant tout sécuriser les investissements publics et privés, sanctionner les opérateurs lorsqu'ils ne respectent pas leurs engagements, renforcer l'ingénierie des collectivités et accroître la transparence et la concertation lorsque des oppositions locales se manifestent. Avant de conclure, j'évoquerai un autre aspect du numérique qui mérite, lui aussi, des investissements à la hauteur : l'illectronisme. En 2020, en France, une personne sur deux n'est pas à l'aise avec le numérique et 13 millions d'entre nous en demeurent éloignés. Si ces inégalités se sont accrues depuis le début de la crise sanitaire, avec le recours parfois indispensable au télétravail, la dématérialisation généralisée des services publics laisse depuis des années sur le bord de la route trois Français sur cinq, incapables de réaliser des démarches administratives en ligne. C'est notamment le cas des personnes en situation de handicap, pour qui 13 % seulement des démarches sont réellement accessibles. L'État a récemment débloqué 250 millions d'euros, en particulier pour le recrutement et la formation de 4 000 conseillers numériques. Dans son rapport, la mission d'information du groupe du RDSE évalue à un milliard la somme à mobiliser d'ici à 2022 pour financer l'inclusion numérique. Loin de nos débats sur le déploiement du très haut débit, ceux qui sont exclus de cette société hyperconnectée ont le sentiment d'être des citoyens de seconde zone. Je vous invite à ne pas les oublier. La

de nos territoires. Quatre demandes sont formulées : l'intégration du très haut débit dans le service universel des télécommunications, la création d'un pôle public des télécommunications, le soutien de l'État dans le financement des réseaux d'initiative publique et le renforcement de mesures plus contraignantes pour les opérateurs privés. Nous sommes néanmoins partagés sur les propositions énumérées dans ce texte, même si l'intention est bonne. Nous souscrivons à l'idée que les réseaux constituent un bien commun, répondant non seulement à des exigences d'universalité, mais aussi de maîtrise de leurs conséquences environnementales. Pour autant, nous nous trouvons actuellement dans une situation de relatif équilibre. Nous pouvons légitimement espérer qu'avec le plan de relance, l'État va accélérer le déploiement de la fibre et veiller à résorber la fracture numérique que connaissent trop de territoires.

La couverture en fibre du territoire national doit indéniablement être totale. Pour autant, possibilité doit être laissée à chacun de choisir son niveau de débit. Je pose la question : tous nos concitoyens ont-ils besoin du très haut débit ? Certes, les périodes de confinement ont pu montrer qu'au sein d'un même foyer, la résilience du réseau pouvait être éprouvée lorsque plusieurs personnes sont connectées en même temps. Néanmoins, à l'heure où la sobriété doit être recherchée, y compris dans le numérique, la mise en place d'un « bon » haut débit peut parfois suffire. Ce serait déjà un véritable saut dans le monde moderne que d'avoir une couverture équilibrée et stable n'excluant plus personne. J'en viens à la question des usages et de l'inclusion numérique, qui me paraît particulièrement importante pour soutenir l'accès de nos concitoyens et de nos entreprises aux outils en ligne. La crise a montré à quel point le développement des usages du numérique était nécessaire, que ce soit pour le télétravail, pour le suivi des cours, mais aussi pour les artisans, pour déposer une demande d'aide auprès de l'État, ou, pour nos concitoyens, pour accéder aux services publics dématérialisés. La mission d'information que nous avons menée au Sénat a cependant montré que près de trois Français sur cinq étaient exclus des usages numériques. Elle préconise entre autres d'évaluer plus finement l'exclusion numérique, de mieux cartographier les zones d'exclusion numérique, de passer d'une logique « 100 % dématérialisation à une logique « 100 % accessible » pour les sites publics en ligne, d'octroyer un crédit d'impôt pour la formation au numérique aux entreprises et en particulier aux PME-TPE, aux commerçants et aux artisans, ou encore de combattre plus efficacement l'exclusion par le coût, avec la création d'un chèque-équipement destiné à la location ou à l'achat d'un équipement de préférence reconditionné, ce qui permet d'ailleurs de servir les objectifs de sobriété numérique en luttant contre l'obsolescence programmée des ordinateurs et des logiciels. Ces propositions nous semblent à même de favoriser la réussite de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, que le Gouvernement a dotée de 250 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. À cet égard, monsieur le secrétaire d'État, je réitère ma question concernant la pérennité de ces financements au-delà des deux ans du plan. En conclusion, le numérique ne saurait se réduire à la seule question de l'aménagement du territoire. Il représente tout un écosystème qui doit contribuer à forger une société société plus égalitaire, sobre et durable. Mais pour atteindre cet objectif, il nous faut rester vigilants sur la stratégie, comme sur le type de réseaux que nous souhaitons déployer. Il faut multiplier les études d'impact, afin de bien mesurer les conséquences de nos choix, avant de les mettre C'est le rôle du politique d'anticiper, d'évaluer les risques et les avantages. Aujourd'hui, aucun domaine n'est cloisonné ; tout est interdépendant. À nous de prendre en compte les multiples dimensions du problème. La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous discutons aujourd'hui d'un sujet ô combien fondamental pour les territoires : l'aménagement numérique. Comme l'ont déjà mis en exergue mes collègues à cette tribune, c'est de fracture numérique que nous parlons aujourd'hui, une fracture qui persiste et qui fait mal ! Au-delà de l'aménagement, il nous faut désormais un plan qui déménage mois de mars 2018, j'avais interpellé le Gouvernement sur l'accès et la qualité des réseaux internet, de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, dont l'état était plus qu'inadmissible dans les territoires, à l'exemple de mon département, le Puy-de-Dôme. La réponse avait été la mise en valeur de la signature d'un accord au mois de janvier 2018, afin d'accélérer la couverture numérique des territoires, qualifiée de plan ambitieux d'inclusion numérique. À cela s'ajoutait l'un des projets pionniers du plan France Très haut débit, avec le déploiement d'un réseau d'initiative publique à l'échelle de l'Auvergne, comme d'autres régions. Malgré quelques améliorations, la situation est loin d'être satisfaisante. La fracture numérique est malheureusement toujours présente ! L'accès au numérique doit rester une priorité partout sur le territoire de la République. La crise sanitaire va bousculer notre mode de vie en matière de mobilité, de lieu de travail et donc d'utilisation du numérique. Comme nous le rappellent les auteurs de cette proposition de résolution, le développement numérique est fondamental pour nos populations rurales qui, comme l'ensemble de la société, vivent une numérisation croissante de leur quotidien, de leur sécurité, de l'accompagnement de leurs aînés et de leur travail. Le développement numérique doit aussi accompagner le retour à la campagne, entamé avec la crise sanitaire de la covid et l'extension du télétravail ; sinon, la fracture numérique va encore s'accroître.

Dans le contexte de la covid, le Gouvernement met en place un plan de numérisation des TPE, dont 30 % seulement disposent d'un site internet, avec une stratégie nationale visant à soutenir la numérisation des petites entreprises. L'objectif est fortement louable : permettre à tous les commerçants, artisans, professionnels de l'hôtellerie et de la restauration de développer une activité en ligne, et ainsi de maintenir leur activité alors qu'ils sont obligés de rester fermés.

que la 5G n'accroisse encore la fracture numérique entre les territoires, si nous ne faisons pas le choix de l'installer sur tout le territoire, ce que je soutiens assurément. Toutefois, aujourd'hui, cela ne semble pas être la solution envisagée : les investissements, sur les cinq prochaines années,

de résolution souhaitent que le service universel des télécommunications intègre l'accès au très haut débit et soit garanti pour tous. Ils s'interrogent sur l'opportunité de créer un pôle public des télécommunications afin de garantir le service universel et la maîtrise publique des infrastructures numériques, notamment de la fibre optique. Ils estiment nécessaire de revoir les architectures de financement des réseaux d'initiative publique afin que l'État accorde un soutien exceptionnel aux collectivités volontaires, au regard de l'importance d'une bonne connectivité pour nos concitoyens. ils souhaitent que des mesures plus contraignantes soient mises en oeuvre afin que les opérateurs privés respectent les obligations qu'ils ont actuellement contractées. En conclusion, pour atteindre son objectif, ce texte étatise fortement le développement numérique et remet en cause l'architecture actuelle. Il ne semble pas nécessaire d'aller si loin. Le tout-État n'a pas fait ses preuves, et, surtout, l'État n'en a pas les moyens - n'en a plus les moyens Les réalisations telles que les réseaux d'initiative publique mises en place par les collectivités locales font leurs preuves. Il faudrait les renforcer. Le temps n'est plus à la recentralisation.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'interviens à la tribune pour la première fois, sur un sujet qui me touche particulièrement, car je suis d'abord une élue de la ruralité. Dans mon village de Gilette, dans les Alpes-Maritimes, comme dans tant d'autres, l'aménagement numérique est une belle promesse à portée de main pour notre avenir. comme les auteurs de la présente proposition de résolution le rappellent, l'accès au numérique peut également engendrer de nouvelles fractures territoriales. Les considérants me semblent donc relever du bon sens.

il semble effectivement difficile de s'opposer à ce voeu pieux. Il est aussi proposé de prendre « des mesures plus contraignantes [ ...] afin que les opérateurs privés respectent [leurs] obligations

Quant à l'exposé des motifs, il me trouble davantage. Quand je lis : « Nous considérons ainsi qu'il est nécessaire de créer un opérateur national, propriétaire des réseaux », franchement, je m'inquiète. Depuis la loi de 2004, nous travaillons pour la confiance dans l'économie numérique, selon un modèle, certes, imparfait. Cela justifie-t-il, pour autant, de remettre en cause tout le travail réalisé par les collectivités territoriales, avec leurs réseaux d'initiative publique ? Franchement, je ne le crois pas.

Monsieur le secrétaire d'État, en revanche, et de façon complémentaire, je m'autorise à revenir sur la place laissée aux collectivités locales de petite taille ou rurales dans le dispositif intéressant leur nécessaire mise à niveau numérique. L'enveloppe de 88 millions d'euros fléchée pour financer la transformation numérique des collectivités locales, sur les 500 millions d'euros prévus pour la transformation numérique du secteur public dans son ensemble, devrait me rassurer. Pourtant, il n'en est rien et je suis préoccupée pour ces collectivités dans le besoin.

Les sillons à géométrie déjà variable du service public s'en trouveront malheureusement plus profonds, selon les territoires. L'État devrait donc leur consacrer plus de temps,

Je rappelle que la France est le seul pays en Europe à avoir fait figurer parmi les critères d'attribution des fréquences 5G une obligation d'équilibre du territoire.

Ceux qui s'opposent à la 5G s'opposeront mécaniquement à la 4G et à la fibre. Il n'y a pas de logique à être pour l'un et contre l'autre. Je reviendrai maintenant sur l'intervention de M. Gontard, que je n'ai pas totalement comprise.

-que nous les avons rassurées à cet égard, notamment sur le caractère simple et opérationnel de l'enveloppe prévue pour les collectivités territoriales. Pour conclure, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai conscience que le déploiement

en application de l'article 50-1 de la Constitution, sur la place de la stratégie vaccinale dans le dispositif de lutte contre l'épidémie de covid-19. Pour l'organisation du débat qui suivra cette déclaration, un temps de parole

ainsi qu'un temps de parole de cinq minutes attribué respectivement à la commission des affaires sociales et à l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il n'y a pas d'observation ? ... Il en est ainsi décidé.